Au nom du Sénat tout entier, je souhaite leur adresser nos vives condoléances pour le drame qu’ils viennent de traverser. Permettez moi également de saluer le professionnalisme et la totale mobilisation des services de secours, notamment les nombreux sapeurs pompiers et gendarmes qui, depuis ce week end, se dépensent sans compter pour rechercher les personnes disparues et pour éviter que d’autres drames ne se produisent. Je pense enfin

Mes chers collègues, par courriers en date des 8 et 11 mars, M. Guillaume Gontard, président du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, et Mme Cécile Cukierman, présidente du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, ont demandé que le projet de loi autorisant l’approbation de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Cambodge, inscrit à l’ordre du jour du jeudi 14 mars, soit examiné selon la procédure normale. Acte est donné de ces demandes. Par courrier en date de ce jour, le Gouvernement a demandé le report de l’examen de ce même projet de loi au mercredi 3 avril, en troisième point de l’ordre du jour. Acte est donné de cette demande.

parlementaire nous a permis de nous mettre d’accord sur la très grande majorité des articles, et même d’y ajouter des dispositifs complétant la protection de l’enfant. Nous avons rendu plus automatique – sans toutefois l’imposer au juge pénal – le retrait de l’autorité parentale en cas de condamnation pour un crime ou une ou une agression sexuelle sur l’enfant ou sur l’autre parent. Par ailleurs, nous avons mis fin au décalage entre le code civil et le code pénal en matière de retrait de l’autorité parentale en introduisant une disposition générale dans le code pénal.

À l’issue des deux lectures successives par nos assemblées, le désaccord portait uniquement sur le régime de la suspension provisoire de l’exercice de l’autorité parentale avant tout jugement.

Toutefois, la commission des lois souhaitait maintenir le principe d’une saisine systématique du juge aux affaires familiales (JAF) par le procureur de la République dans les huit jours pour que la situation de l’enfant puisse être examinée par un magistrat et pour que la suspension ne puisse se prolonger au delà de six mois sans cet examen. Dans notre esprit, c’était là une sécurité pour l’enfant et une manière de vérifier que la mesure était bien appropriée et proportionnée. Le 6 février dernier, le Sénat a finalement adopté la disposition dans la version de l’Assemblée nationale. Il a ainsi accepté que la suspension puisse courir au delà de six mois, tout le temps de la procédure pénale, ou jusqu’à la décision du JAF, lequel serait éventuellement saisi par l’un des parents et non plus systématiquement par le procureur de la République. En revanche, le Sénat a supprimé le régime spécifique de suspension en cas de condamnation, même non définitive, pour des violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail (ITT) de

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, après la belle semaine que nous venons de passer, placée sous le thème des droits des femmes, nous commençons celle ci sous le thème de l’enfance. Vous le savez, la protection de l’enfance constitue, comme celle des femmes, l’une des priorités de notre gouvernement. Aussi, je me félicite que les deux assemblées soient parvenues à un compromis dans le cadre des travaux de la commission mixte paritaire. Il faut dire que le texte que vous avez adopté le 6 février dernier était presque à maturité, puisque seul l’article 1 restait en débat entre l’Assemblée nationale et le Sénat. Cet article, dans la version qui est soumise à votre vote aujourd’hui, modifie l’article 378 2 du code civil afin d’étendre le mécanisme de suspension de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi ou condamné.

à son encontre – jusqu’à la décision de non lieu du juge d’instruction ou la décision de relaxe ou d’acquittement de la juridiction pénale. Certains ont pu penser que cette suspension portait une atteinte

de son désintérêt pour son enfant ; s’il le fait, c’est l’occasion pour lui de démontrer à un juge sa capacité à assurer pleinement le bien être et la sécurité de sa progéniture. L’écriture à laquelle vous avez abouti permet donc d’atteindre nos objectifs de protection de l’enfant en amont de la décision pénale – je ne peux que m’en féliciter. L’article 2, quant a très rapidement fait l’objet d’un large consensus en ce qu’il assure une avancée importante. En l’état du droit positif, le retrait de l’autorité parentale n’est qu’une simple faculté pour le juge, quelle que soit l’infraction ayant donné lieu à la condamnation. Le second volet du dispositif concerne tous les délits commis sur l’enfant à l’exception de l’agression sexuelle incestueuse. En cas de condamnation, le juge pénal aura l’obligation de se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de son exercice. Le troisième Le troisième et dernier volet concerne le cas du parent condamné comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis par son enfant. En cas de condamnation, le juge pénal pourra ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou de son exercice. Je le dis et le redis devant vous ces deux premiers articles constituent une avancée indéniable en matière de protection des enfants. De la même manière que la protection

Aujourd’hui, la France s’engage résolument pour protéger les plus petits d’entre nous. En cela, elle rejoint l’Espagne et l’Italie,

de l’exercice des droits parentaux et qu’elle contraint ou autorise le juge pénal à se prononcer sur le retrait de l’autorité parentale ou de son exercice pour toutes les infractions, de manière proportionnelle à leur gravité. Nous pouvons être fiers de la qualité des travaux parlementaires et des échanges qui ont eu lieu entre les chambres et le Gouvernement. Cela démontre, s’il en était besoin, notre engagement commun au service de la protection de l’enfance. Ce texte, n’en doutons pas, est très attendu par nos concitoyens : parce qu’il renforce la protection des plus vulnérables d’entre nous ; parce que c’est notre devoir de protéger l’enfant victime contre son parent agresseur parce que le foyer doit toujours rester un lieu où l’enfant peut grandir en paix et en sécurité.

Notre groupe a toujours été au rendez vous des avancées législatives acquises en la matière. Tout d’abord, la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste

autonomes sur mineurs de moins de 18 ans dans le cas de l’inceste. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain avait d’ailleurs, par amendement, proposé de relever l’âge du non consentement de 15 à 18 ans dans le cas du crime d’inceste. la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, dite loi Taquet, est venue apporter des améliorations sur les conditions de repérage, d’accueil et d’accompagnement des enfants relevant de la protection de l’enfance. de la protection de l’enfance. Le présent texte prévoit une suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement pour un parent poursuivi ou mis en examen pour crime ou agression sexuelle incestueuse sur son enfant, ou pour crime commis contre l’autre parent pendant toute la durée de la procédure.

Il nous semble donc indispensable de renforcer l’ordonnance de protection. Nous regrettons à cet égard que la proposition de loi de notre collègue Cécile Untermaier, votée à l’unanimité à l’Assemblée nationale le 9 février 2023, n’ait jamais été inscrite à l’ordre du jour du Sénat,

Pour finir sur une note positive, nous tenons à souligner les annonces gouvernementales du mois de mai dernier, notamment la création de pôles spécialisés, qui vont dans la bonne direction.

La protection des enfants fait partie de ces sujets à la fois complexes et sensibles qui nécessitent temps de réflexion, rigueur juridique et travail transpartisan, afin de légiférer de manière efficiente,

Marie Mercier, ainsi que son implication bien connue au sein de cet hémicycle sur les sujets liés à la protection des enfants. La présente proposition de loi met en œuvre plusieurs recommandations issues des travaux de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) et d’associations, dont je salue l’action.

du parent poursuivi pour crime contre l’autre parent ou pour crime ou agression sexuelle commis sur son enfant. L’article 2 pose le principe d’un retrait total de l’autorité parentale en cas de condamnation pour ces infractions. Les chiffres démontrent la nécessité de légiférer. Je n’en citerai qu’un seul, aussi effroyable qu’éclairant : un enfant meurt tous les cinq jours sous les coups de l’un de ses parents. Rappelons que l’autorité parentale est définie par notre code civil comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». Nous savons combien l’autorité parentale est une notion fondamentale en droit de la famille. Le principal sujet de débat entre

le temps de la procédure, c’est à dire jusqu’à la décision du JAF ou celle de la juridiction pénale. Je tiens à saluer ce compromis, convaincue qu’un parent violent ayant commis des crimes sur son conjoint ou sur son enfant ne peut être un bon parent.

essentielle dans la pratique. L’article 2 constitue une avancée indéniable en instaurant l’obligation – et non la faculté – pour le juge pénal de retirer l’autorité parentale ou son exercice en cas de condamnation du parent. Le groupe Les Républicains salue également l’introduction de l’article 2 par la rapporteure, qui prévoit qu’un parent privé de l’exercice de l’autorité parentale par le juge ne peut en demander la restitution avant l’expiration d’un délai de six mois, une fois le jugement devenu irrévocable. ce texte répond à un enjeu particulièrement important : protéger les enfants, faire en sorte que le foyer familial reste un espace de sécurité où l’enfant peut grandir en paix et préserver cette richesse si fragile qu’est l’insouciance de l’enfance. Tel est l’objectif de ce texte ; tel est le souhait que nous partageons collectivement. Je me félicite aujourd’hui que nous y parvenions. La parole

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, les violences intrafamiliales constituent à la fois des drames intimes et un phénomène de masse drames intimes, parce qu’elles brisent la cohésion des familles et chargent les individus d’un immense fardeau ; phénomène de masse, parce que des millions de nos concitoyens ont à en subir les conséquences. On estime en effet que 10 % à 20 % des adultes ont été victimes de telles violences lorsqu’ils étaient mineurs – c’est considérable. Si l’on tient aussi compte de toutes les personnes indirectement concernées par ces violences – les proches, qui ont dû apporter leur aide, mais aussi les associations et les professionnels qui se sont impliqués pour protéger les victimes –, l’on comprend que ces situations concernent une proportion très importante de notre population. Dès lors, comment expliquer qu’il soit si difficile de prendre des mesures fortes pour endiguer ce phénomène ? Précisément parce que les violences familiales, avant d’être un phénomène de masse, constituent des drames intimes. Celui qui commet la violence, parfois le crime, occupe un rôle central dans la structure familiale ; celui là même qui devrait donner de l’amour finit par provoquer de la souffrance. Condamner un parent – le plus souvent un père violent – pour protéger une victime – le plus souvent une mère ou ses enfants – n’est jamais une bonne solution, mais c’est souvent la moins mauvaise. C’est en tout cas celle qui permet de mieux protéger les plus fragiles et d’éviter un engrenage infernal. Le sujet est si délicat qu’il s’avère difficile de prendre des mesures fortes, non par manque de volonté, mais simplement par souci d’équilibre. Après plus d’un an de navette parlementaire, la proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales est sur le point d’être adoptée. Les débats à l’Assemblée nationale et au Sénat ont permis d’aboutir à un texte de compromis.

En première comme en deuxième lecture, notre groupe avait soutenu la position de la commission des lois du Sénat sur l’article 1, qui concentrait l’essentiel du débat. Cet article prévoit la suspension provisoire de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement, dès le stade des poursuites, pour le parent poursuivi pour crime contre l’autre parent ou pour crime ou agression sexuelle commis sur son enfant. Notre groupe jugeait plus pertinent de conserver le caractère temporaire de cette suspension tout en laissant une place centrale au juge dans la procédure. Dans le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire, il n’est plus question du délai maximal de six mois, voté en première lecture par le Sénat. le rôle du juge dans la procédure est renforcé. Nous espérons que cette nouvelle mouture permettra de mieux protéger les enfants : c’est là notre priorité.

Ainsi, la nouvelle version de l’article 1 ne retient plus le cas des violences volontaires ayant entraîné une ITT de plus de huit jours comme motif entraînant la suspension automatique de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement. Cette version nous semble plus équilibrée. Encore une fois, l’objectif est non pas de protéger un parent violent, mais bien de préserver le développement de l’enfant.

400 000 enfants vivent dans un foyer où s’exercent des violences et plus de 160 000 sont victimes chaque année de violences sexuelles. Qu’ils soient directement victimes ou seulement témoins, les conséquences de ces violences

Ce texte va renforcer notre arsenal juridique en permettant, par exemple, de suspendre plus facilement et plus rapidement l’autorité parentale, mais aussi les droits de visite et d’hébergement,

Les droits de la défense, dont il a souvent été question ici, ne sont pas lésés pour autant : le parent concerné pourra saisir le juge aux affaires familiales pour réexaminer un retrait qui aurait été décidé trop vite, ou dans le cadre d’affaires qui traîneraient durant trop longtemps.

Nous savons aujourd’hui qu’elle est fausse et que cette conception de la famille a emporté des conséquences particulièrement douloureuses pour de trop nombreux enfants. Nous savons également, grâce à des témoignages de policiers, que la menace de retrait de l’autorité parentale touche beaucoup de pères. Puissent ils donc réfléchir avant de frapper !

également la suspension du droit de visite et d’hébergement de l’enfant dans le cadre d’un contrôle judiciaire, qui devient le principe et non plus l’exception, comme c’était le cas auparavant.

Nous le savons, la lutte contre les violences intrafamiliales est particulièrement complexe, parce qu’elle touche à l’intime du foyer, mais aussi à certaines conceptions de la société, de la place et du rôle de chacun au sein de la famille. Aujourd’hui, comme nous avons eu l’occasion de le faire à plusieurs reprises ces dernières années, nous faisons un pas de plus dans le bon sens, celui d’une meilleure protection des plus vulnérables. Nous devrions nous revoir prochainement, dans cet hémicycle, afin d’en faire un de plus, avec la création de l’ordonnance de protection immédiate qu’Émilie Chandler et moi même appelions de nos vœux et qui a été votée à l’unanimité la semaine dernière à l’Assemblée nationale. Pas à pas, nous construisons une société plus protectrice pour les femmes, pour les enfants, pour chacun d’entre nous. En conséquence, le groupe Union Centriste votera bien évidemment ce texte.

Ainsi, il a pu mettre son veto à plusieurs procédures, comme le renouvellement du passeport de Paul, qui en avait pourtant besoin pour partir en vacances. En d’autres termes, l’auteur d’un féminicide a conservé l’autorité parentale sur son fils Malheureusement, les cas de l’enfant de Priscilla, de Steffy et de Paul sont loin d’être isolés : 400 000 enfants vivent dans un foyer où se produisent des violences conjugales et 160 000 enfants subissent chaque année des violences sexuelles. Pis, ces enfants sont deux fois victimes, car à la violence physique s’ajoute la violence de la loi, laquelle ne les protège pas entièrement du parent violent. Malgré une attention renforcée, de nombreuses situations ne sont tout simplement pas prévues par les Ces omissions exposent les enfants à un risque inutile et, souvent, à de nouvelles violences qu’un cadre juridique plus protecteur aurait permis d’éviter. La proposition de loi de la députée socialiste Isabelle Santiago – enfant du Val de Marne, tout comme moi – vise justement à construire vise justement à construire un cadre juridique plus protecteur pour les enfants. Pour ne citer qu’un exemple, elle rendrait enfin systématique le retrait de l’autorité parentale en cas de violence sexuelle incestueuse. Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires continue bien évidemment de soutenir ce texte ; nous saluons

lequel l’exercice de l’autorité parentale est suspendu jusqu’à une décision sur le fond lorsqu’un parent est poursuivi par le ministère public pour certaines formes très graves de violences intrafamiliales. Cette suspension est d’autant plus importante que notre système judiciaire reste lent, après des décennies de sous investissement. Le délai de décision au pénal atteignant en moyenne treize mois, des mesures provisoires deviennent indispensables. En parallèle, il faut rendre les métiers de la justice plus attractifs pour permettre des recrutements. En tout état de cause, le compromis trouvé en commission mixte paritaire permet de mieux protéger l’intérêt supérieur de l’enfant. C’est pourquoi nous voterons en sa faveur. Toutefois, ne soyons pas dupes

en œuvre de toute urgence. Nous y veillerons !

l’enfant a le droit au respect de sa dignité et de son amour propre, ne pas piétiner, ne pas humilier, laisser vivre sans décourager, ni brusquer ni presser, du respect pour chaque minute qui passe. Ces mots sont ceux du pédiatre Janusz Korczak, précurseur et inspirateur de la convention des droits de l’enfant. En effet, l’intérêt de l’enfant doit primer : l’enfant doit être protégé à chaque instant de sa vie, et donc tout au long d’une procédure judiciaire le concernant. Cette proposition de loi vise cet objectif, et je nous en félicite, mes chers collègues. S’il a été malheureusement nécessaire de rappeler, durant cette longue procédure législative, que l’intérêt de l’enfant était primordial, le compromis trouvé œuvre en ce sens. Tant mieux ! Tant mieux ! Les chiffres sont édifiants : 400 000 enfants vivent dans un foyer où s’exercent des violences intrafamiliales de manière permanente, et 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles. Ce texte vient donc combler un vide juridique sur la question de l’autorité parentale des parents coupables de violences criminelles et délictuelles sur leurs enfants et sur leurs conjoints.

Tout enfant doit être protégé, y compris de ses parents, quand il le faut. Un parent violent vis à vis de l’enfant ou de l’autre parent ou un parent incestueux ne saurait continuer d’exercer l’autorité parentale non plus que ses droits de visite et d’hébergement. Cette déclaration paraît évidente, elle est désormais légalement automatique. Il est toujours bon de rappeler que l’intérêt supérieur de l’enfant prime sur le droit des parents à influer sur sa vie. C’est bien le parent agresseur qui brise la famille ; il ne peut dès lors que perdre son privilège. Je ne peux que déplorer les nombreux témoignages, recueillis notamment par la Ciivise, de mères séparées s’inquiétant de laisser leur enfant repartir chez un père incestueux, d’un enfant obligé d’aller chez le parent violent en attendant un jugement,

Malgré les avancées législatives de 2019 et de 2020, les enfants ne sont toujours pas suffisamment pris en considération. À ce moment de mon propos, je souhaite saluer le travail remarquable réalisé par la Ciivise, avec à sa tête le juge Édouard Durand,

de stress post traumatique, 50 % des victimes de viol durant leur enfance ont fait une tentative de suicide. Une étude de l’ONU a montré qu’une femme ayant subi des violences physiques et sexuelles dans l’enfance a dix neuf fois plus de risques de subir des violences conjugales et sexuelles à l’âge adulte qu’une femme qui n’a pas vécu ce traumatisme. Un homme qui a connu ce même type de violences a quatorze fois plus de risques d’en commettre à son tour. Suspendre automatiquement l’autorité parentale permettra de protéger l’enfant et l’adulte qu’il deviendra. C’est primordial. Malheureusement, nos enfants ne sont pas que les dommages collatéraux des violences intrafamiliales : ils en sont les victimes. Leur protection doit donc être la plus rapide possible, afin de les mettre à l’abri à limiter tout traumatisme additionnel et à entamer le processus de reconstruction promptement. De plus, ces dispositions permettront de libérer et de protéger la parole des enfants en limitant au mieux les influences perverses de parents criminels cherchant à contaminer leur témoignage.

La balle est désormais dans le camp de l’exécutif pour faire baisser les chiffres édifiants que j’ai cités et pour que la dignité de l’enfant soit préservée. La parole Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, cela fait maintenant plusieurs années que la question des violences intrafamiliales est l’objet d’une prise de conscience

d’entre nous, je me réjouis que la navette arrive enfin à son terme concernant cette proposition de loi et je tiens à une nouvelle fois à saluer ses auteurs ainsi que notre rapporteure, Marie Mercier. Nous avons souvent eu l’occasion de travailler ensemble au sein de la commission des lois et je connais son implication sur ces sujets.

importantes. Ainsi, l’article 2 établit le principe d’un retrait total de l’autorité parentale en cas de condamnation pour crime commis sur l’autre parent ou d’agression sexuelle incestueuse ou crime commis sur l’enfant. J’ai également à l’esprit différents enrichissements du texte initial, comme l’exonération de toute obligation d’informer préalablement l’autre parent d’un changement de résidence en cas d’ordonnance de protection.

le contenu a déjà été rappelé en détail. Cet article introduit une suspension provisoire de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale en cas de poursuites pour crime commis sur l’autre parent ou de crime ou agression sexuelle commis sur l’enfant et en cas de condamnation pour violence conjugale. Le groupe RDSE a pris position en deuxième lecture, avec un amendement déposé par notre collègue Nathalie Delattre. Nous étions en accord avec l’Assemblée nationale, même si nous entendions les avertissements de notre rapporteure.

À titre personnel, je considère que nous n’aurions pas dû avoir peur d’aller plus loin, mais la démocratie et le parlementarisme imposent à chacun une culture du compromis comme du consensus.

Un samedi soir, fin septembre, Lisa a été battue à mort. Son corps portait de multiples hématomes d’âges différents sur le visage, le thorax, le dos, le pubis et les quatre membres. Ce drame effroyable fut largement relayé par la presse nationale. Ses bourreaux exerçaient depuis plusieurs années des violences répétées sur Lisa et sur son frère de 6 ans

Le chemin législatif de ce texte a été long. J’admets être soulagée que les sénateurs et les députés membres de la commission mixte paritaire soient parvenus à un accord,

marque une avancée essentielle dans la protection de l’enfance : il faut protéger le plus tôt possible les enfants victimes de ces violences ; leur mise à l’abri est une nécessité urgente et impérieuse. Tous les cinq jours, un enfant est tué par l’un de ses parents ; plus d’un infanticide est commis chaque semaine dans notre pays. Ces chiffres sont édifiants.

Comme l’a rappelé notre collègue députée Isabelle Santiago, auteure de cette excellente proposition de loi, un parent agresseur ou violent ne peut être un bon parent : la seule boussole est l’intérêt supérieur des enfants.

le crime ou l’agression sexuelle incestueuse contre l’enfant parmi les motifs de suspension automatique des droits parentaux. Ce manquement est comblé par le présent texte. Ainsi, nous pouvons espérer que les enfants victimes ou covictimes de violence seront plus facilement extirpés des situations dangereuses

judiciaire. Cette disposition est cohérente avec le reste des articles que nous avons déjà votés conformes. Elle s’inscrit dans la même ambition de protection de nos enfants, dans le prolongement des travaux qui ont été menés depuis le Grenelle des violences conjugales en 2019.

aux voix l’ensemble de la proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire. Mes chers

La séance est reprise. L’ordre du jour appelle discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à faciliter la mise à disposition aux régions du réseau routier national non concédé (proposition n° 347, texte

la loi 3DS a introduit la possibilité d’une mise à disposition de parties du réseau routier national non concédé, à titre expérimental, aux régions volontaires. En cela, cette loi, construite dans la concertation et le dialogue avec les élus et leurs associations, constitue une innovation par rapport aux précédents actes de décentralisation routière elle ne prévoit pas un classique transfert aux départements comme par le passé, mais offre la possibilité aux autorités organisatrices des mobilités à l’échelle régionale de prendre la main sur la gestion, la modernisation et l’aménagement des axes routiers les plus structurants de leurs territoires. Trois régions – Occitanie, Auvergne Rhône Alpes et Grand Est – ont saisi l’opportunité et se sont portées volontaires pour s’engager dans cette démarche, concernant un linéaire total de plus de 1 600 kilomètres de routes et d’autoroutes. Les régions Grand Est et Auvergne Rhône Alpes ont d’ores et déjà conclu avec l’État une convention de mise à disposition entrant en vigueur au 1 janvier 2025. Les discussions sont en bonne voie avec la région Occitanie pour finaliser la mise au point de la convention. Le conseil régional doit se prononcer le 28 mars Les régions candidates ont toutefois unanimement relevé une lacune dans le texte adopté en 2022, qui compromet, voire empêche l’exercice des nouvelles missions des régions en l’état, au vu de la jurisprudence claire et constante du Conseil d’État, les présidents de conseil régional ne sont pas habilités à déléguer leur signature aux agents de l’État. Or quiconque est familier de la gestion d’un réseau routier sait la quantité d’actes administratifs et réglementaires qui sont nécessaires au quotidien. Chaque direction interdépartementale des routes (DIR) sera ainsi amenée à émettre chaque année des centaines d’arrêtés de circulation pour travaux, interventions ou gestion d’événements sur la voie publique, des centaines, voire des milliers, de bons de commande pour réparer, entretenir, maintenir le patrimoine routier, et autant pour en exécuter la liquidation – et cette énumération Les services aguerris à la gestion des routes, qu’il s’agisse de ceux de l’État, des départements ou des métropoles, sont ainsi dotés de chaînes de délégations de signature qui permettent au niveau le plus pertinent d’agir avec réactivité au bénéfice des usagers de la route. La présente proposition de loi permettra de transposer la même fluidité dans l’action au quotidien dans le cadre des expérimentations régionales, en précisant le périmètre de compétence du président du conseil régional et en autorisant les délégations et les subdélégations vers les directeurs et les agents des services de l’État.

en instaurant une possibilité de délégation de signature du président du conseil régional au service de l’État mis à la disposition de la région pour la gestion du réseau routier confié dans le cadre de l’expérimentation.

loi Maptam, a fait des régions les chefs de file pour l’exercice de la compétence mobilité. La loi 3DS du 21 février 2022, votée quelques années plus tard, a complété ce dispositif en matière de mobilité, en permettant le transfert définitif de routes aux départements et la mise à disposition, aux régions volontaires et à titre expérimental, du réseau routier national non concédé. Cette expérimentation doit durer huit ans et s’achever en 2030.

À l’issue de l’adoption de la loi 3DS, les régions Grand Est, Auvergne Rhône Alpes et Occitanie ont manifesté leur souhait de bénéficier de l’expérimentation. Le 4 janvier 2023, le ministère des transports a indiqué à ces trois collectivités locales les autoroutes et routes nationales qu’il entendait mettre à leur disposition, un total de 1 638 kilomètres. Après cette décision, les négociations entre l’État et les régions se sont poursuivies pour procéder à la signature d’une convention encadrant cette mise à disposition.

En effet, l’article 40 de la loi 3DS, qui prévoit l’expérimentation, ne permet pas au président de région de déléguer sa signature aux agents de l’État. Or le code général des collectivités territoriales ne prévoit pas non plus que le président du conseil régional puisse déléguer, de manière générale et en toute matière, sa signature à des agents de l’État. Le Conseil d’État est particulièrement vigilant sur ce point : il n’hésite pas, par exemple, à sanctionner les délégations de signature du conseil départemental à des agents de l’État dépourvues de base légale.

Tout au long de l’expérimentation, même si les régions délèguent en pratique leur signature aux services de l’État pour la signature des actes administratifs du quotidien, ce sont bien les régions qui prendront toutes les décisions de gestion, d’investissement et d’aménagement des routes mises à leur disposition. L’État ne prendra donc plus aucune décision concernant les routes mises à disposition jusqu’à la fin de l’expérimentation. À mon sens, le texte adopté par la commission est complet et ne pose aucune difficulté technique ou juridique. Les services du ministère des transports m’ont du reste indiqué que la proposition de loi répondait

car son rejet conduirait inévitablement à une gestion totalement inefficace des routes transférées. Oui, il convient de permettre aux régions candidates d’assurer le bon exercice de la compétence nouvelle dont elles vont disposer.

Ces blocages seraient du reste préjudiciables à l’entretien, à la rénovation, à la modernisation de ce réseau transféré, dont l’état n’est déjà pas extraordinaire, faute d’une attention suffisante de la part de son gestionnaire.

À ce jour, on peut surtout évoquer une fragmentation accrue de la compétence routière, exercée par les communes et les intercommunalités sur 700 000 kilomètres de route,

Je ne conteste pas le chef de filât des régions en matière de mobilité. Je souligne simplement que les départements y apportent leur part, notamment pour ce qui concerne les infrastructures routières de proximité.

la faute à un État central qui asphyxie méthodiquement et toujours davantage un échelon départemental pourtant d’une grande utilité pour répondre aux attentes de nos concitoyens.

en outre judicieux, dans le cadre de la seconde vague de mise à disposition annoncée, de revisiter les conditions du transfert que beaucoup ont considérées, à juste titre, comme constitutives d’un marché de dupes.

ses dimensions territoriales.

Les pluies incessantes et les inondations qui en résultent, les forts gels ou encore les canicules malmènent nos routes et provoquent des dégradations prématurées. Le manque d’entretien et de moyens

français. Les solutions sont multiples. Je partage l’idée que la subsidiarité dans ce domaine est primordiale. Les différentes strates, État et collectivités territoriales, proposent un panel de réponses. Organiser leur articulation doit conduire à des changements concrets et à une amélioration

J’ai également entendu votre engagement, monsieur le ministre, à discuter des meilleures solutions avec notre assemblée. Nous répondrons bien entendu présents, tant le sujet est d’importance. Nous devons être guidés par le bon sens et la recherche de solutions logiques et pragmatiques.

son rapporteur, l’excellent Alain Marc. Le rapport a été très largement soutenu, ce qui prouve que lorsque l’on constate un obstacle et que l’on opte pour une solution réaliste et efficace, cela a du sens.

qu’un transfert appelle non pas une simplification des règles, mais un complément législatif. Nous examinons aujourd’hui la proposition de loi visant à faciliter la mise à disposition aux régions du réseau routier national non concédé.

sur la question des départements ruraux et des transferts de routes nationales. L’objectif de ce texte est de combler un oubli de nature technique et, partant, de faciliter l’application de l’article 40 de la loi du 21 février 2022, la fameuse loi 3DS.

la région Grand Est, qui aura notamment la possibilité d’expérimenter l’écotaxe gérée par la région, la région Auvergne Rhône Alpes et l’Occitanie. Le ministre des transports a formalisé les portions de route mises à leur disposition en tout début d’année 2023,

actuellement géré par les DIR et les Dreal, force est de constater que l’État n’est plus en mesure d’entretenir le réseau national. Il a en effet perdu des compétences indispensables et se montre incapable de décliner ses propres engagements relatifs au réseau routier national dans les contrats de plan État région

contrer les reports de trafic de transit. Combinée avec la taxe analogue que prépare la Collectivité européenne d’Alsace sur son périmètre propre, elle incitera à l’optimisation logistique et au report modal tout en tout en dégageant des moyens pour accompagner la décarbonation des véhicules et les investissements routiers de modernisation. Cette mise à disposition s’inscrit dans un mouvement de décentralisation des routes engagé depuis une cinquantaine d’années au moins,

Cette expérimentation régionale sur des axes majeurs est gage d’une mise en œuvre pertinente et territorialement adaptée de la transition écologique des mobilités, que ce soit par l’instauration de voies dédiées aux cars express et aux bus à haut niveau de service, par des aménagements favorisant l’autopartage ou par le déploiement de bornes de recharge électriques. La possibilité offerte aux régions de conduire l’aménagement d’axes stratégiques en cohérence avec leur politique de transition des mobilités permettra indéniablement d’accélérer et d’amplifier l’efficacité de l’action publique. Il est donc utile que la région, si elle en a la volonté, puisse prendre la main sur ces axes dans le cadre d’une politique de transport adaptée et cohérente pour le territoire. Pour y parvenir, il faut toutefois en avoir les moyens.

les collectivités territoriales, notamment les régions, subissent un contexte financier défavorable qui n’est sans doute pas étranger au fait que seulement trois régions aient opté pour cette expérimentation. Nous sommes loin d’un formidable engouement régional.

des chaînes de délégation depuis le président de l’exécutif régional jusqu’aux agents sur le terrain. Le groupe écologiste votera bien évidemment pour cet ajustement législatif.

On peut donc dire qu’il n’y a pas eu un grand enthousiasme de la part des collectivités à reprendre une partie du réseau national, ce qui ne doit pas nous surprendre.

pourrait conduire à soumettre certains itinéraires aux aléas et caprices des différentes autorités de transport qui auraient à s’en occuper. On ne peut exclure que, pour certains itinéraires reliant un point A à un point B, l’usager de la route ait à traverser des portions appartenant à plusieurs institutions différentes, qui n’auront pas toutes forcément la même approche des politiques routières. Nous aurions tout de même besoin d’une cohérence nationale pour structurer notre réseau national… La présente proposition de loi prévoit que, sur demande des régions volontaires pour la reprise de fractions du réseau routier national,

Tout cela intervient dans un contexte où les négociations sur les modalités financières des transferts n’ont pas abouti et où les négociations des contrats de plan sont toujours en cours. Il aurait pu être intéressant de profiter de cette occasion pour proposer des financements complémentaires aux régions.

entre l’État et les régions. Les présidents de région seraient ainsi habilités à signer des documents pour les fractions de route nationale continuant à relever pour partie de la compétence de l’État. Avouons qu’il s’agit tout de même d’une curieuse modalité de décentralisation ! Au moment du vote de la loi 3DS, je ne suis pas sûr que nous avions prévu une telle différenciation ni une simplification aussi compliquée. Même si la procédure consistant à passer par une nouvelle proposition de loi pour résoudre un problème juridico administratif apparaît comme la seule solution,

nous ne voulons pas non plus nourrir un blocage contre les exécutifs des régions qui ont eu l’audace de se lancer dans cette aventure et qui devront l’assumer. C’est pourquoi nous nous abstiendrons.

En l’état actuel du droit, la possibilité pour l’exécutif régional de déléguer sa signature à des agents de l’État mis à disposition ne peut être mobilisée pour l’exercice d’une compétence transférée ou mise à disposition. En outre, le droit ne permet qu’une délégation aux chefs de services déconcentrés alors que, pour la gestion des routes, des subdélégations au sein même des services sont nécessaires.

l’Occitanie, le Grand Est et Auvergne Rhône Alpes. Celles ci vont donc récupérer à titre expérimental la gestion de 1 638 kilomètres d’autoroutes et routes nationales pour une période de huit ans. l’on compte les départements et les métropoles parties prenantes de l’expérimentation, près de 30 % du réseau routier national ont changé de main

il n’est pas surprenant que nous ayons à ajuster le tir pour satisfaire les exigences du Conseil d’État, alors que les conventions ne sont pas encore toutes signées. Il s’agit surtout de rendre effective dans les meilleurs délais l’expérimentation prévue pour les régions.

En commission, nous avons considéré que cette proposition de loi n’avait pas à être modifiée compte tenu de l’objectif visé. Néanmoins, les membres du groupe RDSE voteront

qui vise à rendre pleinement opérationnelle l’expérimentation permise par la loi 3DS du 21 février 2022. Cette loi a ouvert la voie, à titre expérimental pour une durée de huit ans, à la délégation de la compétence d’aménagement et de gestion des routes nationales et autoroutes non concédées concédées aux régions volontaires. Je tiens à rappeler le caractère précurseur, en matière de différenciation, de la Collectivité européenne d’Alsace. Celle ci s’est en effet vue transférer, au moment de sa création, la propriété des routes et autoroutes non concédées,

conformément à la loi Maptam. Cette expérimentation répond par ailleurs à une demande de l’association Régions de France qui, dans un contexte de dégradation du réseau concerné, proposait en 2017 que l’exercice de la compétence soit confié aux régions. Actuellement, trois régions se sont engagées dans cette voie et les modalités de l’expérimentation sont en cours de finalisation. Il convient de saluer le caractère novateur de ces transferts, qui illustre aussi bien la dynamique de décentralisation et de différenciation voulue par le Président de la République que la capacité d’innovation des collectivités territoriales. Ce sont les régions volontaires qui définissent, en partenariat avec l’État, les modalités de l’expérimentation sur leur territoire. Elles disposent ainsi d’une certaine liberté dans la manière dont elles pourront gérer

Quant aux régions Auvergne Rhône Alpes et Occitanie, elles en ont profité pour assumer plus efficacement leur qualité de chef de file en matière de mobilité. Plus concrètement, le texte que nous examinons vise à lever certains obstacles pratiques au déploiement concret de cette expérimentation sans en altérer l’esprit ni les

que l’État est censé mettre à leur disposition pour l’exercice de ces compétences. Aussi, afin de ne pas fragiliser le bon déroulement de l’expérimentation, l’article unique de cette proposition de loi complète utilement l’article 40 de la loi 3DS en permettant précisément au président du conseil régional, et éventuellement aux personnes à qui il a délégué son pouvoir, de donner délégation de signature aux agents de l’État intervenant sur le réseau routier mis à disposition.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi s’inscrit dans une trajectoire de modernisation nécessaire au bon fonctionnement de notre réseau routier.

La loi 3DS, en autorisant l’expérimentation du transfert aux régions volontaires de la compétence d’aménagement et de gestion des routes nationales et autoroutes non concédées, poursuit cette évolution.

Cette expérimentation, entreprise par les régions Grand Est, Occitanie et Auvergne Rhône Alpes, a révélé des difficultés techniques et opérationnelles, en particulier lors des négociations entre les régions et l’État. Résoudre les défis identifiés par les régions concernées, tel est l’intérêt du texte En effet, la relation entre l’État et la région est l’un des moteurs de l’action publique qui permet aux collectivités territoriales de poursuivre leur effort de territorialisation. Si le réseau non concédé représente seulement 1,1 % du réseau routier national, il n’en est pas moins stratégique en ce qu’il concentre 19 % du trafic routier.

Comme vous le savez, une lacune majeure a été identifiée : les actions quotidiennes relevant des attributions de pouvoir adjudicateur et d’ordonnateur, en matière de gestion et de conservation des infrastructures routières, requièrent une délégation de signature aux services et agents chargés des réseaux routiers fournis par l’État. Ce texte vient combler cette faille technique. Les modifications apportées lors des débats à l’Assemblée nationale, notamment l’allongement du délai de huit à seize mois pour la négociation des conventions de mise à disposition des routes, démontrent une volonté d’adapter le texte aux réalités du terrain. Cela semblait essentiel pour éviter tout litige juridique en cas de dépassement du délai initial et pour sécuriser juridiquement les opérations à venir. de répondre à une demande légitime des régions, qui cherchent à assumer pleinement leurs responsabilités en matière d’aménagement du territoire. Cependant, à ce jour, force est de constater que cette expérimentation n’a pas suscité l’enthousiasme tant attendu. C’est

mais sans esprit de contrainte, tel est l’objet de ce texte. En outre, il aurait pu être pertinent que la convention de mise à disposition entre l’État et la région précise le périmètre exact du domaine et des installations concernés, le but étant de clarifier les négociations qui interviennent après la décision ministérielle, afin de définir finement les voies, routes et autres biens inclus dans ce périmètre. Les régions restent des entités républicaines créées par les lois de décentralisation de 1981. Il est fondamental de garantir et de faire évoluer leurs libertés.

Cette proposition de loi fait suite aux transferts successifs des routes aux collectivités territoriales. En effet, le réseau routier national s’amenuise d’année en année. De par une évolution progressive, notamment l’acte II de la décentralisation, qui a transféré aux départements les deux tiers du réseau routier national, on compte désormais à peine plus de 11 000 kilomètres de routes nationales non concédées contre 37 000 kilomètres de routes départementales. Pour sa part, la loi 3DS du 21 février 2022 en ses articles 38 et 40 permet aux départements et aux métropoles de récupérer un certain nombre de routes. Dans le même temps, l’article 40 introduisait, à titre expérimental pour huit ans, une procédure de mise à disposition de certains axes du réseau routier national non concédé par l’État aux régions volontaires. Cette mise à disposition temporaire n’a séduit que trois des treize régions métropolitaines : le Grand Est, l’Occitanie et Auvergne Rhône Alpes.

Cette demande était justifiée par les fortes contraintes de circulation sur cet axe et par un nombre très élevé d’accidents. Dans sa réponse à l’État, le département fixait néanmoins trois conditions suspensives, à savoir savoir un état des lieux précis de l’intégralité des charges transférées, notamment pour le personnel, une compensation de l’État pour les charges nouvelles excédant les charges de fonctionnement et d’investissement ordinaires et l’engagement de l’État de contribuer, au moins pour 50 %, au programme de modernisation de l’itinéraire financé par le contrat de plan État région. Sur cette demande, le département s’est vu opposer une fin de non recevoir au motif que « le calcul d’une compensation financière liée à la décentralisation, constitutionnellement garantie, ne peut donner lieu à une négociation spécifique entre l’État et la collectivité territoriale bénéficiaire du transfert

Elle répond à un véritable besoin des trois conseils régionaux concernés par les transferts expérimentaux de routes nationales. Je ne veux pas revenir sur le fond du texte, car mes collègues l’ont déjà très bien fait, notamment Pierre Alain Roiron.

Comme en 2021, je considère que pour que ces expérimentations soient des succès, il faut définir les modalités les plus adéquates au cas par cas, avec les acteurs concernés, et les mettre en cohérence avec les besoins qui peuvent être ceux des régions intéressées. Dès lors qu’elles n’ont été que trois à se lancer, j’estime que la loi 3DS est partiellement en échec. Aussi avais je songé à déposer un amendement visant à rouvrir la possibilité pour les régions de demander des transferts, qui auraient conservé le caractère expérimental, mais en différenciant, décentralisant et déconcentrant véritablement les négociations des contrats entre l’État et les régions – c’est à dire en étudiant chaque projet individuellement, tant j’estime que la durée fixe de huit ans n’est pas transposable à chaque réalité locale et à chaque projet. La région Grand Est, qui est la seule à pouvoir instaurer une écotaxe, a besoin de ressources financières importantes pour amortir les investissements lourds et nécessaires sur les axes transférés expérimentalement, à commencer par l’élargissement et le verdissement de l’A31. Mais il a fallu attendre dix huit mois pour que l’ordonnance écotaxe soit publiée : autant de temps et de ressources perdus pour la région, alors même qu’elle doit en parallèle travailler avec les directions interdépartementales des routes pour parfaire le partage de l’expertise technique, et avec les conseils départementaux pour agir de concert face aux risques de fuite des poids lourds sur les axes voisins de l’A31. Plus généralement, une incertitude pèse sur l’effectivité des compensations financières liées à ces transferts : celles ci sont régies par les contrats de plan État région or les nouveaux volets mobilité desdits contrats s’étendent sur la période allant de 2023 à 2027. Ils ne couvrent donc pas l’intégralité de la durée de ces expérimentations, entre 2022 et 2030, et ne permettent pas aux conseils régionaux concernés de mener des politiques ambitieuses sur ces réseaux. Je sais que les régions attendent ce texte. Je n’ai donc pas déposé d’amendement pour ne pas risquer de compromettre l’adoption conforme. Monsieur le ministre, pouvez vous nous dire si vous êtes prêt à relancer des cycles d’expérimentations de transferts en modifiant l’article 40 de la loi 3DS et, cette fois ci, en renforçant en renforçant les volets budgétaires et temporels comme je viens de l’indiquer ? Avant de lancer des conventions citoyennes sur les mobilités, n’oublions pas de régler d’abord les tracasseries du quotidien par des textes pas assez bien écrits ni préparés, ce qui oblige les parlementaires, en l’occurrence David Valence, député de votre majorité, à devoir rectifier le tir Le groupe socialiste votera en faveur de ce texte court, précis et utile pour nos collectivités régionales. S’il vous plaît, monsieur le ministre, et à travers vous c’est à tout le Gouvernement que je m’adresse, travaillons autrement sur le volet législatif et écoutons davantage

Aux termes de plusieurs décrets précisant les modalités et compensations de ces transferts, la situation est aujourd’hui celle d’un partage possible entre départements, régions et métropoles pour la gestion par les régions des routes nationales et des autoroutes non concédées.

Lors de l’examen de la loi 3DS au Sénat, le 8 juillet 2021, nous avions initialement supprimé l’article qui permettait à l’État de transférer des routes du réseau national aux régions volontaires. Le second élément que je voudrais évoquer concerne le rôle de l’État. La loi 3DS a ouvert la troisième phase de désengagement de l’État dans le réseau routier, après des transferts massifs aux départements en 1972 et 2006. Aujourd’hui, quel rôle l’État

L’État a concédé ce tronçon restant à réaliser au département de l’Aveyron. L’engagement financier substantiel de ce département et de la région Occitanie montre la volonté de faire avancer ce projet d’intérêt national.

Ce dossier aveyronnais expose la complexité actuelle de la gestion du réseau routier principal par les collectivités territoriales et l’État. Pour revenir plus directement au texte que nous examinons, cette proposition de loi est technique, comme l’ont rappelé

chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat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

La séance est reprise. L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi,

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, le texte dont nous débattons cet après midi

J’ai entendu les préoccupations de nos agriculteurs qui se trouvent de plus en plus souvent confrontés à des néoruraux souhaitant s’installer au vert sans en accepter toutes les conséquences. Je le dis, cela n’est pas acceptable. Si l’on choisit la campagne,

j’ai fait connaître ma volonté d’avancer sur cette question, afin de faire cesser les procès ubuesques que l’on voit fleurir régulièrement. Car, oui, notre campagne est un milieu vivant, parfois même bruyant odorant, un milieu dans lequel des femmes et des hommes se lèvent tôt, travaillent avec passion et sans compter leurs heures, pour nous nourrir. Derrière les affaires qui peuvent prêter à sourire, on cherche à faire taire le coq Maurice ou les cloches d’une église, il y a des situations humaines, des enjeux économiques, qui méritent que l’on s’y attarde. des actions en justice, parce qu’elles sont incommodées par le bruit des moissonneuses batteuses.

le respect absolu de ceux qui vivent et travaillent chez eux depuis toujours. Qu’il me soit permis d’insister ici sur un élément qui, je le crois, sera un point clé lors de nos débats : si ce texte répond à un besoin réel de nos campagnes, il a vocation à s’appliquer à toutes les relations de voisinage, puisque nous créons un nouvel article dans le code civil. de la même manière les voisins des villes comme les voisins des champs. Je pense, par exemple, à la pizzeria du rez de chaussée qui, certes, dégage des odeurs et est bruyante, mais qui était là avant que de nouveaux habitants n’emménagent au premier étage. La proposition de loi consacre tout d’abord le principe jusqu’alors jurisprudentiel de la responsabilité fondée sur les troubles anormaux de voisinage : chacun a le droit de jouir paisiblement de sa propriété, de son logement, de son fonds et a droit à réparation du préjudice qu’il subit. C’est ce principe simple, partagé par tous, qui est repris dans le présent texte. Il s’agit d’une responsabilité sans faute. L’introduction de ce principe général dans le code civil le rend plus lisible et accessible ; elle renforce la sécurité juridique du droit français et assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi. devant la loi. Le texte institue par ailleurs une exception générale tirée de la théorie dite « de la pré occupation », afin de trouver un meilleur équilibre entre les différents intérêts en présence. est, mesdames, messieurs les sénateurs, le cœur du sujet qui nous occupe, car cette disposition fixe le principe selon lequel celui qui s’installe à proximité d’un lieu particulièrement bruyant ou polluant ne peut se plaindre d’un trouble anormal du voisinage, alors même que la nuisance existait au moment de son installation.

L’exception a ainsi été étendue à celui qui exerce son activité dans des conditions nouvelles si celles ci ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble. est de ne pas limiter à l’excès les possibilités d’évolution des activités en question, de ne pas les figer dans un carcan qui limiterait leur développement, tout en les encadrant, pour ne pas nuire excessivement au voisinage.

économiques » à la notion d’activités, afin de préciser le type d’activités visées par l’exonération. Vous avez également précisé la notion d’« installation de la victime sur les lieux ; vous avez ainsi privilégié la référence à un acte juridique en identifiant « l’acte ouvrant le droit de jouissance de la personne qui allègue subir le dommage Permettez moi cependant d’exprimer une réserve sur ces modifications, qui restreignent le champ d’application du texte.

le plus général possible et à englober tous types d’activités, de quelque nature qu’elles soient. De la même manière, la référence à « l’acte ouvrant le droit de jouissance » paraît trop restrictive et difficilement compréhensible. En effet, cette rédaction, contrairement à celle de l’article L. 113 8 du code de la construction et de l’habitation – dont elle s’inspire n’inclut ni l’obtention d’un permis de construire ni la conclusion d’un acte authentique de vente, ce qui limite significativement la portée de l’exonération de responsabilité.

dans le cas où le trouble anormal provient d’activités nouvelles résultant d’une mise en conformité de l’exploitation. Seront examinés tout à l’heure des amendements tendant et de la pêche maritime, afin de satisfaire le souhait de nos agriculteurs de bénéficier d’une protection plus forte lorsque l’exercice de leur activité évolue. Cette préoccupation est légitime ; le Gouvernement y est particulièrement sensible. Nous devons cependant rester attentifs dans la suite de nos débats

d’égalité des citoyens devant la loi, ainsi que du droit à un recours effectif. Ne perdons pas de vue notre objectif

engagées contre des agriculteurs par des voisins quérulents, qui se plaignent de nuisances liées à leur activité. L’odeur du bétail, le bruit des tracteurs, le chant du coq ou encore le meuglement des vaches poussent certains de ces nouveaux habitants à saisir la justice, à l’instrumentaliser et à s’opposer à des exploitations qui étaient là bien avant leur arrivée. que décourager les recours contentieux, ce texte doit également servir d’instrument de dialogue entre voisins et contribuer à trouver une solution amiable,

que la tentative de médiation ou de conciliation préalable à la saisine du juge s’applique précisément aux troubles anormaux de voisinage. Je forme le vœu

puisse contribuer, dans le droit fil de la politique de l’amiable, à la pacification des relations de voisinage sur l’ensemble du territoire et au désengorgement des tribunaux. C’est en somme

odeurs de bétail, la pollution visuelle due à une cheminée d’usine ou de simples nuisances provoquées par des voisins irrespectueux, les troubles anormaux de voisinage font partie du quotidien de nos concitoyens.

l’application de la cause exonératoire de responsabilité, dès lors que la modification des conditions d’exercice de l’activité

à l’extension à diverses activités de la cause exonératoire, la commission a relevé l’indétermination relative de la notion et les difficultés d’application qu’elle pourrait poser : doit on vraiment exonérer

ouvrant le droit de jouissance de la personne qui allègue subir le dommage », notion qui présente le double avantage de prévoir une datation précise et de renvoyer à une réalité juridique plus objective et conforme au principe selon lequel « celui qui vient aux nuisances ne peut s’en plaindre La discussion aura à nouveau lieu sur ce point, mais nous avons cherché à faire œuvre utile en précisant des notions qu’à défaut il appartiendra à la jurisprudence de circonscrire, avec les aléas et les incertitudes que cela emporte. nous avons souhaité compléter la codification de la jurisprudence qu’opère la présente proposition de loi, en prévoyant les conditions, actuellement déterminées par la jurisprudence, dans lesquelles le juge judiciaire peut, cas d’une activité autorisée par l’administration, ordonner des mesures visant la réduction ou la cessation du trouble anormal de voisinage. Nous avons tenu compte à cet égard de la jurisprudence du Tribunal des conflits, qui a émis des réserves sur la compétence du juge judiciaire en la matière,

régulièrement, les médias attirent notre attention sur des contentieux liés à des troubles de voisinage en milieu rural, en raison du mode de vie à la campagne ou des activités agricoles. Le son des cloches de l’angélus, le chant du coq, le bruit des tracteurs et des moissonneuses batteuses, les odeurs à proximité d’exploitations agricoles, le meuglement des vaches, le bêlement des brebis : oui, la ruralité a ses spécificités liées aux diverses nécessités du travail agricole et à la vie villageoise. S’ils peuvent prêter à sourire tant ils apparaissent cocasses, anecdotiques ou semblent reposer sur des motifs futiles, ces litiges traduisent parfois des situations très complexes. L’anormalité de ces troubles de voisinage est appréciée par le juge qui se fonde sur une jurisprudence abondante. La proposition de loi que nous examinons cet après midi a pour objet de moderniser et de compléter le droit de la responsabilité civile en insérant dans le code civil un volet relatif aux conflits de voisinage. Elle consacre ainsi une jurisprudence bien établie, afin que le principe de responsabilité fondée sur les troubles anormaux de voisinage à la campagne, comme à la ville, puisse être appliqué à l’ensemble du territoire de manière uniforme. Une exception à ce principe est néanmoins prévue par le texte. En effet, le juge peut écarter cette responsabilité, dès lors que le trouble résulte d’une activité qui est à la fois préexistante préexistante à l’installation du nouveau voisin et conforme à la législation en vigueur, et que cette activité s’est poursuivie dans les mêmes conditions après l’installation du nouvel arrivant. Ces trois conditions cumulatives garantissent ainsi un juste équilibre entre les intérêts de chacun.

de cette mise en conformité. Je me réjouis de l’insertion de cette précision. Avant de conclure, je tiens tout particulièrement à saluer l’action de médiation et de conciliation des maires des petites communes rurales. En effet, ils œuvrent avec dévouement et abnégation à l’apaisement des relations de voisinage entre les ruraux et les nouveaux arrivants lorsqu’un désaccord surgit. Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, cette proposition de loi, en apportant

Elle permettra de réduire les conflits de voisinage, en protégeant notamment nos agriculteurs contre les actions abusives intentées par certains nouveaux habitants des territoires ruraux.

d’origine sénatoriale par le passé. Ce texte s’inscrit dans un travail plus large d’adaptation de la responsabilité civile aux enjeux actuels. Comme cela a été évoqué à de nombreuses reprises au cours de nos travaux, la responsabilité civile – ou l’obligation pour chacun de répondre du dommage causé à autrui et d’en assumer les conséquences

Aussi ne peut on que se réjouir de légiférer pour mieux encadrer ce droit, qui est le fondement de notre vie en société, la base de notre capacité à cohabiter.

L’inscription dans le code civil du régime de la responsabilité civile pour troubles anormaux de voisinage a été souvent envisagée, mais toujours repoussée. On ne peut donc que féliciter notre collègue de l’Assemblée nationale

interpellés et sollicités pour résoudre les troubles de voisinage. Il en va de même pour les préfets, les procureurs, les juridictions, alors que l’on dénombre près de 18 000 dossiers ayant trait à un trouble anormal du voisinage. Bien entendu, certaines de ces plaintes sont sans fondement

Plus globalement, nous considérons que cette proposition de loi, qui codifie la jurisprudence, est indubitablement la bienvenue, dans un contexte de judiciarisation croissante des problèmes de voisinage. Le dispositif proposé est clair et équilibré et la clause exonératoire, fondée sur la théorie de la pré occupation et ses trois critères – respect de la législation, antériorité du trouble et poursuite, dans les mêmes conditions, de l’activité qui en est à l’origine – est empreinte de réalisme. Enfin, si nos débats portent sur une proposition de loi, pour répondre aux troubles anormaux de voisinage, n’oublions pas la prépondérance des liens sociaux et des relations de proximité à l’échelle du quartier : bien souvent, ils demeurent les meilleurs remèdes aux maux humains. C’est bien lorsque toutes les modalités de dialogue et de conciliation ont été épuisées que cette loi doit s’appliquer. Mes chers collègues, je vous confirme, car vous l’aurez compris, que le groupe Union Centriste votera cette proposition

Cette notion juridique, consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation, s’appuie sur l’appréciation du juge au fond, qui, seul, détermine la nature du trouble – bruits, odeurs, Elle est caractérisée, comme l’a rappelé la rapporteure, par l’existence d’un dommage, l’anormalité du trouble, la relation de voisinage entre le défendeur et le demandeur, selon l’appréciation du juge.

considèrent que ces dispositions établissent vis à vis du premier occupant une « servitude légale de pollution », tendant à « pérenniser les situations nuisibles à l’environnement

serait limitée ou sanctionnée au prétexte d’un préjudice visuel. Cette différenciation nous semble inégalitaire. Nous regrettons ce réarmement juridique qui, encore une fois,

emporter des conséquences très importantes sur des contentieux qui impliquent des exploitations agricoles polluantes – qui seraient, par exemple, passées d’un élevage moyen à un élevage intensif – ou des activités industrielles.

Loin de se limiter à une structuration juridique nécessaire, le texte se drape dans une défense qui nous paraît caricaturale de la ruralité et de l’agriculture qui serait perturbée et empêchée par l’arrivée des rats des villes.

de ceux qui analysent l’explosion des litiges entre voisins comme le symptôme d’un climat social dégradé et d’un affaiblissement du lien social dans notre pays. C’est vrai ! Bien souvent, les premiers remparts contre ces phénomènes sont les collectivités locales : les maires et les autres élus locaux endossent le rôle – souvent ingrat, il faut bien le dire – de médiateurs et de conciliateurs pour tenter, tant bien que mal, d’y faire face. Il reste que les troubles de voisinage sont la cause de querelles et d’actions judiciaires qui pourrissent le quotidien d’un trop grand nombre de foyers, en ville comme à la campagne.

Tout acteur déjà installé n’aurait donc plus à réparer les dommages qu’il pourrait causer à son nouveau voisin du fait de son activité. Cette rédaction déniait tout droit de recours à une partie de la population victime d’un trouble anormal de voisinage et créait, en quelque sorte,

nous voterons ce texte.

les conflits de voisinage augmentent et, quand la zizanie s’installe, l’ensemble de la collectivité en pâtit. Dans ma commune de Damazan, dont j’ai eu l’honneur d’être le maire pendant quinze ans, j’ai bien sûr connu ce type de conflits délicats, notamment lors de la création d’entreprises.

Préserver l’harmonie d’un lieu signifie non seulement préserver le cadre de vie et le droit de propriété des citoyens, mais également protéger nos entreprises, qui font vivre nos territoires. Si l’intitulé ambitieux de cette proposition de loi peut paraître en décalage avec son dispositif, qui se limite à un pan spécifique de la responsabilité civile, les questions abordées relèvent au fond de sujets majeurs pour la ruralité. Il est proposé de consacrer dans le code civil un régime de responsabilité prétorien pour les dommages causés par les troubles de voisinage dits anormaux. Si l’on trouve la première mention de ces troubles dès 1844, conséquence de la révolution industrielle et de la mutation de nos modes de vie, de consommation et de production, le législateur s’est tenu éloigné de cette question. Le juge judiciaire a ainsi construit un régime autonome du droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle disposé dans le code civil. Qualifié de souple, ce régime laisse au seul juge la faculté d’apprécier le critère de gravité de la nuisance, au cas par cas.

Pour en revenir au texte qui nous occupe, je tiens d’abord à saluer le travail de Mme la rapporteure. Très bien ! Si les principes de la jurisprudence établie sont conservés, la limitation de la cause exonératoire aux seules activités économiques bouleverse l’équilibre qui a été trouvé à l’Assemblée nationale.

ailleurs, je souligne la prévoyance de notre commission, qui a tenu à remédier à l’imprécision de la notion d’« installation » et à préserver la compétence de l’administration – donc du juge administratif – pour les troubles autorisés par elle.

C’est oublier que la ruralité, avant d’être un espace de repos ou de loisir, est un espace de production artisanale et industrielle, tout particulièrement agricole.

En effet, bloquer le développement d’une exploitation au niveau d’activité qui existait au moment de l’installation d’un nouveau voisin, c’est la condamner. Une exploitation qui ne peut pas se développer, c’est une exploitation qui ne peut pas s’adapter aux évolutions et aux besoins du secteur.

Dans le même esprit, pour protéger encore davantage les activités préexistantes, nous défendrons également un amendement visant à étendre la protection contre les recours abusifs aux activités non économiques. Le principe général serait ainsi le suivant : celui qui choisit de s’installer, en toute connaissance de cause, à proximité d’une source de nuisances, quelle qu’en soit la cause, économique ou non, ne peut pas engager une procédure fondée sur les troubles anomaux de voisinage.

d’une société contemporaine qui prône le respect de l’autre et le vivre ensemble, mais qui, pourtant, butte au quotidien, voire se fracasse sur les délicats accommodements entre les hommes, sur la cohabitation parfois douloureuse de l’homme et de son environnement ou encore sur la difficile conciliation de la vie humaine avec les activités économiques, agricoles ou commerciales. Cette proposition de loi a donc pour objectif ambitieux de contribuer à apaiser cette cohabitation,

les collectifs de riverains qui ne sont pas convaincus après la tentative de médiation iront au contentieux. Ils ne gagneront peut être pas toujours, d’autant moins si la charge de la preuve leur incombe désormais au premier chef, mais ils se est ce vraiment donner sa meilleure chance au vivre ensemble dans notre pays, dans nos villes et dans nos campagnes que de voter une proposition de loi qui ne convainc pas pleinement ? N’est ce pas, au contraire, contre productif ? Ne serait il pas préférable de continuer de faire œuvre pédagogique en nous appuyant sur la subtile expertise des juges

sont aussi de plus en plus exigeants quant à leur liberté individuelle et à leur bien être ou confort personnel. En somme, cette proposition de loi révèle une autre facette d’un phénomène déjà bien connu : le Nimby. Tout le monde Tout le monde est pour les panneaux solaires, les bornes de tri, les bancs publics, les logements sociaux, la campagne nourricière, les bistrots du coin, mais personne ne les veut trop près de chez soi, trop près de son jardin, trop près de sa cour.

en paradis sur terre. On aura beau faire le procès des néoruraux qui ne s’accommodent pas de leurs voisins agriculteurs, seront ils plus conciliants si on les renvoie en ville, là où l’on prône la densification pour éviter l’étalement urbain ? Qui plus est, si l’on ne répond pas aux angoisses des urbains, quand on refait la ville sur la ville, où iront ils, si ce n’est dans le périurbain ou le rural ? Au fond, ne partons nous pas un peu trop du principe que tous ces voisins râleurs, futurs ou actuels, auraient le choix de leur habitation Je ne reviens pas sur la crise immobilière ou sur la pénurie généralisée de logements abordables. Dans nos villes comme dans nos villages, on n’a pas franchement le privilège de pouvoir choisir son voisin et son voisinage… Les Français les plus aisés, oui ; les autres – et ils sont majoritaires –, rarement.

Demander à de futurs occupants de se renseigner de manière plus précise sur l’environnement de leur futur chez soi, à l’aide des notaires par exemple, est évidemment pertinent, mais, je le répète, cela ne vaut que pour ceux qui ont véritablement le choix. C’est rarement le cas du demandeur d’un logement social, de l’étudiant qui cherche une chambre ou du salarié qui ne veut pas être trop éloigné de son emploi

Tenir compte du déjà là, faire avec le déjà là : ces expressions et démarches sont appréciées des architectes et urbanistes qui pensent la ville durable. Nous y souscrivons pleinement. Parfois, nous devons protéger le déjà là : c’est notamment le rôle des défenseurs du patrimoine, que celui ci soit architectural, sensoriel, vert ou autre. Parfois, nous devons au contraire ne pas figer le déjà là, mais l’enrichir – étendre un bâtiment, agrandir une ferme, surélever un immeuble ou bâtir en fond de parcelle.

Aussi, parce que les associations de locataires se montrent manifestement réservées, même sur le texte issu de notre commission des lois, parce que des membres du Conseil national du bruit ont exprimé leur opposition,… Ils l’ont fait bruyamment… … parce que les collectifs de riverains, urbains comme ruraux, continuent de s’interroger sur l’utilité de modifier nos codes, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises, nous avons en effet besoin de clarifier encore la situation pour répondre notamment à l’inquiétude des organisations agricoles. Cela passe par l’inscription dans le marbre de la loi d’une adaptation de la responsabilité civile aux enjeux actuels, car nous sommes encore trop souvent témoins de recours abusifs de nombreux voisins à l’encontre d’agriculteurs. Aussi, l’Assemblée nationale a proposé la rédaction d’un nouvel article 1253 du code civil civil définissant le principe de la responsabilité « de plein droit » de certaines personnes « à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage », rédaction à laquelle a été ajoutée une clause exonératoire de responsabilité s’appliquant lorsque le trouble anormal causé à la personne lésée provient d’activités, quelle que soit leur nature, préexistantes à son installation, qui se sont poursuivies dans les mêmes conditions et sont conformes aux lois et règlements. Rappelons qu’actuellement la notion juridique de « trouble de voisinage » n’existe pas dans le code civil. Pour s’adapter aux changements de vie de notre société, un régime de responsabilité particulier et autonome a été progressivement créé par le droit jurisprudentiel. De ce fait, il revient au juge d’apprécier et de manière objective l’anormalité du trouble en question.

l’antériorité du trouble, l’adaptation à la législation en vigueur et la poursuite de l’activité, qu’elle soit agricole, industrielle, artisanale, commerciale, touristique, culturelle ou aéronautique. Dans ce contexte juridique, un arrêt de la Cour de cassation de 2023 a considéré que, dans un village

en ce qu’elle ne se concentrait pas sur les activités économiques et qu’elle ne prenait pas suffisamment en compte les spécificités liées aux activités agricoles. Elle a donc apporté des précisions spécifiques aux conditions d’application de ce texte à ces mêmes activités agricoles.

postérieurement à l’acte ouvrant le droit de jouissance de la personne qui allègue subir le dommage, dans des conditions nouvelles résultant de la mise en conformité de l’exercice de ces activités aux lois et aux règlements ». Il apparaît en effet anormal qu’un exploitant agricole puisse être condamné pour trouble du voisinage, alors qu’une disposition législative ou réglementaire viendrait l’obliger à modifier les

chers collègues, un certain nombre d’associations ou de collectifs représentant les victimes de troubles de voisinage se sont inquiétés du risque que la rédaction du texte issu de l’Assemblée nationale faisait peser sur le principe de trouble anormal de voisinage. En effet, il était initialement prévu que la clause exonératoire s’appliquerait dès lors que ce trouble proviendrait d’activités, « quelle qu’en soit la nature ». Cette formulation trop imprécise privait le juge de toute marge d’appréciation et risquait d’empêcher des recours susceptibles d’être véritablement justifiés. Rappelons que l’objectif de ce texte est aussi de mieux protéger les citoyens des effets néfastes liés aux troubles de voisinage. La version sénatoriale du texte semble donc mieux répondre aux inquiétudes exprimées par nos agriculteurs, en leur offrant un environnement juridique plus sûr et plus visible.

mettre fin à la judiciarisation excessive, pour ne pas dire abusive, liée à la surréaction de certains néoruraux, d’autant plus quand ces troubles ont précédé ont précédé l’installation de ces nouveaux arrivants. Même s’il sanctuarise particulièrement les activités agricoles, ce texte renforce la sécurité juridique du droit français et conforte plus généralement le droit de chacun de nos concitoyens à pouvoir jouir paisiblement de son bien.

le régime de responsabilité pour troubles anormaux de voisinage. Ce régime, dégagé dès le milieu du XIX siècle par la jurisprudence, et affiné depuis, prévoit, pour reprendre la formulation de la Cour de cassation, que « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ». Le législateur est néanmoins d’ores et déjà intervenu pour encadrer ce régime, qu’il a inscrit dans le code de la construction et de l’habitation, en l’accompagnant d’une clause exonératoire de responsabilité en cas de pré occupation, c’est à dire dans le cas où une activité causant un trouble anormal préexiste à l’installation du voisin demandeur. Il s’agit là d’une conciliation nécessaire entre le droit à la quiétude, d’une part, et les nécessités de l’activité économique, d’autre part.

L’une des manifestations de cette crise est sans nul doute le sentiment de rupture du lien entre le monde agricole et une partie des Français. En témoigne la multiplication dans les journaux des affaires de contentieux

bucolique de la campagne, et les agriculteurs qui confère au présent texte une forte actualité. Cependant, bien que le Premier ministre une adoption rapide de ce texte comme élément de réponse à la crise agricole, je n’identifie pas, à l’issue des travaux de l’Assemblée nationale, de dispositifs nouveaux de nature à prévenir l’inflation contentieuse dont sont victimes nos agriculteurs : pas un amendement du Gouvernement à l’Assemblée nationale ni même au Sénat

Je salue à ce titre l’amendement adopté en commission des lois, sur l’initiative de sa rapporteure, qui prévoit, au sein du code rural et de la pêche maritime, une clause exonératoire spécifique à l’agriculture, relative aux troubles résultant d’une mise en conformité de l’exploitation. Comment imaginer qu’un agriculteur ait à choisir entre se conformer aux nombreuses normes en vigueur et s’exonérer de sa responsabilité ? Néanmoins, je considère qu’il reste possible de pousser le curseur un cran plus loin, dans le respect du droit au recours effectif, pour prévenir les contentieux résultant de la vie normale d’une exploitation, notamment de l’évolution de ses activités ou de son agrandissement. Pourquoi un jeune agriculteur qui s’installe avec soixante vaches, pour débuter dans le métier, ne pourrait il pas, comme tout entrepreneur souhaitant développer son activité, dégager du revenu et amortir le coût de ses investissements

de textes précédemment déposés ici, au Sénat, mais aussi des réflexions du Conseil d’État, pour une meilleure sécurisation des activités agricoles. Très bien ! Il y a là, monsieur le garde des sceaux, de quoi véritablement revenir vers le monde agricole en lui disant : voilà ce que nous avons fait pour vous ! Du concret, du concret, encore du concret : voilà ce qu’attendent nos agriculteurs. Ne manquons pas l’occasion, par ce texte, de leur en donner. La parole est à M.

je m’interroge sur l’approche retenue et sur ses implications potentielles. Je tiens à souligner que, dans un contexte où la modernisation de notre droit est une nécessité, nous devrions aspirer à une réforme qui intègre de manière cohérente l’ensemble du droit de la responsabilité civile. L’exemple de L’exemple de la Belgique, qui a récemment entrepris une révision globale de ce droit, nous montre qu’une modernisation exhaustive et réfléchie est non seulement possible, mais également bénéfique. L’accent mis par la proposition de loi sur une facette particulière du droit de la responsabilité civile, sans tenir compte de la complexité et des nuances des relations de voisinage, soulève des questions importantes. En adoptant une vision plus large, englobant à la fois le droit de la responsabilité civile et le droit des biens, nous pourrions parvenir à une compréhension plus nuancée et à des solutions plus adaptées à la diversité des situations que nos concitoyens rencontrent

des conséquences juridiques, nous risquons en effet de laisser place à une incertitude qui pourrait affaiblir l’efficacité de la réforme et miner la confiance dans notre système législatif. Il est impératif que nous nous cette lacune, pour nous assurer que la législation apporte une réponse adéquate et juste à ceux qu’elle cherche à protéger. Il est également essentiel de souligner que notre objectif commun est de trouver des solutions pragmatiques qui répondent aux besoins réels de notre société, sans précipitation ni partialité. Dans cette optique, cette proposition de loi pourrait constituer un premier pas vers une réforme plus complète et équilibrée, qui saura tenir compte des enjeux actuels. Une telle démarche nous permettrait de répondre de manière plus adéquate aux besoins de tous les secteurs de notre société, en tenant compte spécifiquement des défis posés par la crise agricole qui viennent d’être évoqués. Vous me permettrez de citer un défi que nous devrions affronter prochainement, celui du « zéro artificialisation nette » (ZAN), puisque les experts ne cessent de nous alerter sur l’explosion des troubles

Par cet amendement, il est proposé de revenir au texte de l’Assemblée nationale, pour ne pas limiter son application aux seules activités économiques.

Il me semble en effet extrêmement important d’appliquer à l’ensemble des activités le principe de responsabilité civile pour troubles anormaux du voisinage et de ne pas limiter ce principe aux seules activités économiques. Je partage également votre proposition de suppression de la notion d’« acte ouvrant le droit de jouissance ». Cette notion ne permet pas de faire référence de manière claire

Mercier. Monsieur le président,

l’environnement – du régime des exonérations de responsabilité pour trouble anormal de voisinage. Ces installations répondent à un régime d’autorisation environnementale spécifique prévu aux articles L. 511 1 A à L. 511 2 du code de l’environnement, car elles peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage. En l’espèce, l’article unique prévoit d’exonérer de responsabilité les activités agricoles et les activités économiques qui bénéficient de la théorie de la pré occupation.

Le régime d’exclusion de responsabilité prévu par le texte pourrait, dans certains cas, heurter le principe du droit d’agir en responsabilité et, plus généralement, celui du droit au recours effectif, en privant les victimes d’un trouble anormal de toute possibilité juridictionnelle de le faire cesser.

présenter l’amendement n° 1 rectifié. Cet amendement a pour objet d’exclure de la catégorie des troubles anormaux de voisinage les effets sonores causés par les enfants dans les services aux familles, les aires de jeux pour enfants et les installations similaires. petite enfance, dite Norma, l’espace extérieur est obligatoire dans toutes les nouvelles crèches situées dans un kilomètre carré accueillant moins de 10 000 habitants et fortement recommandé dans les autres établissements. Pour autant, de nombreuses crèches subissent des conflits de voisinages, les habitants à proximité de ces établissements considérant que les enfants font trop de bruit. Concrètement, les crèches concernées peuvent faire face à des refus de mise à disposition de l’usage des espaces communs au droit du local de la crèche, des refus d’autorisation d’aménagement des espaces communs à usage privatif, aménagements pourtant exigés par la réglementation relative à la protection des enfants, et des restrictions d’usage des espaces communs par une copropriété, contraires aux intérêts des enfants. Pour garantir leur liberté individuelle et favoriser leur épanouissement, il me semble important de consacrer un droit des enfants à faire du bruit.

Je vous remercie

Nous espérons sincèrement que les débats au Sénat permettront la mise en œuvre du droit effectif des enfants à faire du bruit. Trop de crèches, victimes de conflits de voisinage, se voient

on doit accepter que, pendant un temps limité, dans un espace dédié, des enfants puissent jouer et se défouler – ce qui ne fait pas de nos enfants des barbares. La mise en œuvre de la théorie jurisprudentielle du trouble anormal de voisinage a pu déboucher sur la condamnation de collectivités – je fais ici vécues –, sur le fondement d’éléments objectifs, au motif que les enfants pouvaient faire du bruit dans une cour de récréation le matin, l’après midi et au cours de la pause méridienne. Cet amendement tend donc à élargir la clause exonératoire, ce qui permettra de prévenir ce type de contentieux pour le moins abusif et d’éviter que les collectivités qui sont chargées de la gestion et du fonctionnement de ces établissements scolaires ne soient traînées en justice par des riverains nouvellement installés, sous prétexte que les enfants font du bruit. Quel

Pour autant, il ne s’agit évidemment pas de permettre tout et n’importe quoi. C’est la raison pour laquelle nous nous référons à la notion de « modification substantielle » : la limite posée à l’agriculteur serait une modification substantielle de son activité et des nuisances

d’une exonération de responsabilité lorsque son activité a connu une modification non substantielle. Prenons l’exemple d’un élevage de chiens qui passerait de vingt à vingt

les conditions de son exploitation pourra bénéficier d’une exonération de responsabilité s’il démontre qu’il n’en résulte pas pour son voisin

telle disposition revient en réalité à exonérer l’exploitant auteur d’un trouble anormal de voisinage qui aurait fait évoluer de manière substantielle ses conditions d’exploitation, au motif que la nature ou l’intensité du trouble n’a pas été substantiellement modifiée. Cette rédaction, selon le Gouvernement, revient à priver la victime du trouble de tout droit à réparation, alors qu’elle a subi une aggravation de son dommage. Or on ne peut refuser d’indemniser un préjudice au seul motif que celui ci n’est pas substantiel. Cela va d’ailleurs à l’encontre du principe de réparation intégrale du préjudice en droit de la responsabilité civile.

la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à lutter contre les discriminations par la pratique de tests individuels

la lutte contre les discriminations est bien évidemment une ardente nécessité. Notre gouvernement est profondément engagé à promouvoir l’égalité sous toutes ses formes dans la société, ce qui implique un combat résolu et sans relâche contre toute discrimination. Malgré l’inscription formelle de l’égalité dans nos textes fondateurs, la réalité montre que cet idéal est encore loin d’être atteint pour nombre de nos Il devient donc impératif d’assurer à chaque individu l’accès mérité à des opportunités d’emploi, à un logement décent, ainsi qu’aux prêts bancaires nécessaires pour concrétiser ses projets personnels ou professionnels.

Cette réalité est encore plus prégnante au sein des communautés issues de l’immigration, où 82 % des individus rapportent avoir été discriminés, principalement en raison de leur origine ou de leur couleur de peau. Nous ne pouvons vivre avec ces constats. Les domaines de l’emploi et

telle résignation témoigne d’un profond désespoir. Cette proposition de loi vise précisément à redonner espoir à ces Français, en leur offrant les moyens de se défendre et de réclamer justice.

Ce mécanisme implique l’envoi de candidatures fictives, différenciées par des critères susceptibles d’être discriminants, afin de recueillir des données permettant d’analyser les pratiques discriminatoires à grande échelle et d’identifier les organisations fautives.

en effet la réalité objective. Ce texte, largement révisé par la commission des lois du Sénat, a pour ambition de fournir aux victimes de discrimination un véritable parcours judiciaire. Le Gouvernement, par voie d’amendement, exprimera sa volonté de réintroduire les articles supprimés en commission, car il considère que leur suppression met en péril l’esprit initial de la proposition de loi. Il nous faut pouvoir fournir aux acteurs publics des outils reconnus, afin de faire évoluer les comportements et de lutter efficacement contre les discriminations.

La proposition de loi prévoit également la création d’un comité des parties prenantes, qui réunirait des parlementaires, des experts et, évidemment, le représentant du Défenseur des droits. Cette structure aura pour mission de choisir

exemple – afin d’évaluer si elles ont toutes les mêmes chances de prospérer. Si tel n’est pas le cas, on est en présence d’une situation de discrimination potentielle. La méthodologie des tests serait élaborée en concertation avec un comité des parties prenantes, rassemblant pêle mêle des parlementaires, des experts ainsi que des représentants des organismes susceptibles d’être testés, des employeurs, des salariés et des associations – tel était l’objet en second lieu, de prévoir une procédure de suivi spécifique aux tests statistiques. Celle ci s’appuierait sur un dialogue entre l’État, la Dilcrah, le comité des parties prenantes, ainsi que l’administration du travail. De manière générale, l’organisme épinglé serait soumis à une obligation de négociation en vue de conclure un accord portant sur des mesures correctives ou, à défaut, d’établir unilatéralement un plan d’action.

Si la commission des lois a largement remanié la proposition de loi, ce n’est pas en raison d’un quelconque désaccord sur le constat. Ne nous voilons pas la face, les discriminations existent ce domaine, le combat est loin d’être gagné. Je rappelle que la Défenseure des droits a reçu plus de 6 700 réclamations en matière de discrimination en 2023, contre 5 215 en 2021. Les trois principaux critères sont le handicap, pour 21 %, l’origine, pour 13 %, et l’état de santé, pour 9 %. Ces chiffres sont plus que préoccupants et nous partageons tous pleinement la volonté de lutter contre les discriminations. Hélas ! la qualité d’une loi ne se mesure pas à ses bonnes intentions… C’est vrai ! … et nous avons considéré qu’en l’espèce le dispositif proposé n’était pas la voie la plus adéquate pour lutter efficacement contre les discriminations. Je ne m’attarde pas sur la question de la nécessité d’une intervention du législateur pour parvenir aux objectifs visés – chacun se fera son idée. Sur le fond, l’examen de la proposition de loi en commission a démontré que plusieurs de ses dispositions étaient imprécises, incomprises, voire franchement contre productives. Je pense tout d’abord aux tests individuels de discrimination. La proposition d’en confier la réalisation à la Dilcrah a, je dois le dire, fait l’unanimité contre elle.

Nous avons fait droit à leurs arguments : la Défenseure des droits nous est bel et bien apparue comme l’institution la plus pertinente pour assurer cette mission. Elle dispose d’une expertise de longue date en la matière et est la mieux placée pour accompagner les victimes dans la suite de la procédure, y compris en cas de contentieux. Concrètement, elle dispose de pouvoirs d’enquête et peut recourir à la voie de la médiation, émettre une décision portant recommandation ou, en cas de contentieux, produire des observations devant le juge. Enfin, son indépendance est une plus value indéniable dans les cas où une personne publique est en cause. Afin de ne pas créer de concurrence entre les acteurs de la lutte contre les discriminations – une telle concurrence ne profiterait à personne, surtout pas aux victimes –, nous avons donc entendu préserver la compétence de la Défenseure des droits sur ce point. En conséquence, nous avons limité la compétence de la Dilcrah à la seule réalisation de tests statistiques. J’en viens à l’article 2 et au comité des parties prenantes. Celui ci a été présenté par l’auteur de la proposition de loi comme le moyen de prévenir toute critique quant à la robustesse de la méthodologie des tests. Je rappelle qu’une grande campagne de tests statistiques a été conduite par l’État en 2019 2020, mais que cette initiative n’a pas pu prospérer du fait de critiques particulièrement vivaces émises par les entreprises épinglées à l’encontre de la méthodologie employée. Il serait illusoire de penser que la création d’un énième comité permettrait de couper court aux contestations. Il serait également naïf d’imaginer que toutes les entreprises se rallieraient à la cause du simplement parce que la loi le leur prescrit. Au fond, on cède ici à la tentation bien française de vouloir tout régler par la création d’une nouvelle norme… Le comité des parties prenantes nous est apparu d’autant plus inadapté que les modalités concrètes de son fonctionnement, notamment sur la majorité requise, Autant l’unanimité semble hors de portée compte tenu de sa composition, autant une mise en minorité des entreprises ouvrirait d’entrée de jeu la voie à des contestations. Ce format est en outre excessivement rigide. Afin de favoriser l’émergence d’un consensus, il apparaît plus pertinent de laisser aux pouvoirs publics la liberté d’établir au cas par cas le format d’échange le plus adapté, étant entendu que les partenaires sociaux devront systématiquement y être associés. Enfin, les missions dévolues à ce comité feraient de lui bien plus qu’un conseil scientifique, puisqu’il interviendrait à de nombreuses reprises dans la procédure de correction des pratiques faisant suite à un test statistique. Si les résultats d’un test statistique laissent présager de pratiques discriminatoires, il revient pourtant en priorité à l’administration du travail d’accompagner l’entreprise pour qu’elle mette en place, en concertation avec les représentants du personnel, des mesures correctives.

J’en viens maintenant au cœur du réacteur, à savoir l’article 3, qui a trait aux suites apportées aux tests statistiques. Je voudrais être très claire sur ce point : nous ne sommes pas opposés à la mise en place de campagnes de tests statistiques par l’État.

Correctement utilisés, les tests s’inscrivent donc dans une démarche vertueuse. En revanche, ils ne doivent pas être pris pour ce qu’ils ne sont pas et il serait imprudent de faire d’un instrument avant tout statistique l’alpha et l’oméga de la lutte contre les discriminations. Je rappelle qu’un test ne permet de détecter que certaines catégories de discrimination dans un laps de temps déterminé. Comme toutes les études sur le sujet le rappellent, ces tests ne révèlent qu’un fragment des pratiques des organisations et ne permettent pas de tirer des conclusions définitives quant à d’éventuelles discriminations. Ces rappels méthodologiques étant faits, j’en viens à l’épineuse question des suites apportées aux tests de discrimination. L’article 3 prévoyait une procédure particulièrement insatisfaisante, et ce pour trois raisons. raison porte sur sa complexité, voire son illisibilité. La procédure pouvait se découper en une dizaine d’étapes, pas toujours clairement articulées, et durer jusqu’à deux ans. En des temps de sobriété normative, il y avait de Sur le fond, elle comportait également deux vices majeurs : d’une part, l’absence de phase contradictoire préalable permettant de purger les situations où une entreprise apporte des réponses convaincantes aux anomalies détectées ; d’autre part, le risque d’interférence, que j’ai déjà évoqué, entre le comité des parties prenantes et le dialogue social interne à l’entreprise. La deuxième raison a trait à la philosophie de la procédure qui, comme trop souvent en la matière, n’a d’autre finalité que la sanction : cette approche ignore les initiatives déjà prises par les entreprises, par exemple dans le cadre des négociations obligatoires – un accord national interprofessionnel a été conclu en 2006 et l’on observe un foisonnement d’accords au niveau des branches. Je pense aussi aux outils de droit souple, par exemple le label diversité, ou à l’auto auquel ont recours certaines entreprises, comme le groupe Casino. Les sanctions prévues me laissent d’ailleurs dubitative l’efficacité du fait l’objet de nombreux débats sans qu’aucun consensus émerge, tandis que l’amende administrative risque fort de ne pas être appliquée. La troisième raison est aussi la plus importante : le droit du travail nous offre déjà tous les instruments nécessaires. Rien n’empêche un dialogue informel entre l’administration du travail et une entreprise visée par un test. Si l’accompagnement bienveillant a parfois ses limites, l’État est toutefois loin d’être désarmé quand il s’agit de répondre aux entreprises les plus récalcitrantes. L’inspection du travail dispose d’une compétence générale pour contrôler l’application des dispositions du code du travail et, le cas échéant, engager une action en recherche des discriminations, voire saisir le parquet.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous avons supprimé l’article 3. Mes chers collègues, gardons nous de confondre une juste cause avec une bonne loi. La commission des lois a trouvé un équilibre satisfaisant autour d’un triptyque simple

l’une de nos valeurs fondamentales, inscrite à l’article 1 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Nous considérons que seul le mérite doit fonder les distinctions entre les individus. Cet idéal politique étant au cœur de notre pacte républicain, nous nous félicitons qu’il soit toujours objet de consensus. Main dans la main avec le droit, dans le cadre d’une concurrence loyale et non faussée, l’économie de marché contribue à réduire les discriminations. Le développement du capitalisme s’est accompagné d’une réduction majeure des discriminations économiques infligées à des groupes religieux, raciaux ou sociaux particuliers. Milton Friedman nous rappelle t il que la « main invisible » d’Adam Smith ne distingue pas selon l’origine ou l’appartenance réelle ou supposée des individus. Elle ne distingue pas et elle ne doit pas distinguer il y va d’un principe d’efficacité économique, qui profite tant aux individus qu’à la société dans son ensemble. Non seulement les discriminations gâchent la vie de ceux de nos concitoyens qui y sont confrontés, mais elles freinent également le développement de notre économie. rapport de France Stratégie indique que nous perdons chaque année plusieurs points de croissance en raison des discriminations qui perdurent dans notre pays. Nous n’avons donc aucune excuse, mais nous avons de solides raisons politiques et économiques pour lutter activement contre les discriminations. Il ne suffit pas, hélas ! de décréter l’égalité en droit pour qu’elle devienne réalité. Il nous faut lutter constamment contre les discriminations qui portent atteinte à cet idéal. Dans notre droit, du reste, la discrimination est un délit puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Ces peines sont bien entendu renforcées en cas de circonstances aggravantes. En dépit de cette sévérité, force est de constater que de telles pratiques perdurent. Le sentiment de discrimination progresse même parmi nos concitoyens, singulièrement parmi nos concitoyennes. Le texte que nous examinons aujourd’hui a vocation à améliorer notre droit la création d’un service destiné à détecter les pratiques discriminatoires par la réalisation de tests. Il prévoit également une procédure permettant de sanctionner les manquements constatés. Ces objectifs sont louables ; le dispositif envisagé se heurte malheureusement aux efforts déjà déployés pour lutter contre les discriminations. Le Défenseur des droits est en la matière un acteur majeur et il réalise déjà des tests individuels dont l’objet est de mettre en évidence les discriminations.

La procédure de sanction prévue à l’article 3 a également été supprimée en commission, eu égard aux outils déjà présents dans notre arsenal juridique. Nous soutenions bien entendu le caractère plus pédagogique d’une démarche qui visait à compléter l’approche répressive.

qu’elles se généralisent. Nous ferions mieux de continuer à renforcer les moyens de la justice, pour lui permettre de traiter efficacement ces affaires : seuls nos tribunaux garantissent efficacement le droit à un procès équitable. de loi nous permettra de mieux comprendre le phénomène discriminatoire et, par conséquent, de mieux lutter contre celui ci. Nous devons continuer de veiller à faire reculer les différences de traitement, les inégalités et les discriminations dans notre pays.

plus de 6 700 réclamations ont été formées en 2023, contre 5 200 deux ans plus tôt – encore cette augmentation alarmante ne traduit elle pas toute l’ampleur réelle du phénomène. Les chiffres relatifs aux catégories les plus discriminées ne sont que les révélateurs de la mobilisation des associations qui accompagnent les réclamants. Saluons leur rôle essentiel, tant il est vrai qu’il est difficile de convaincre les personnes victimes de discrimination d’aller devant le juge. Reste que la photographie statistique n’est pas réaliste. Je veux me

La couleur de peau, le genre, l’orientation sexuelle, l’âge, la religion, l’engagement politique ou encore le handicap : l’énumération des motifs qui poussent un être humain à en écarter un autre est aussi longue que douloureuse.

Cependant, nous devons veiller à ne pas nous doter d’outils redondants ou d’organismes concurrents. Gardons nous de l’affichage comme du déni ! Aussi, je veux saluer le travail précieux réalisé par la commission des lois, en particulier par notre rapporteure, Catherine Di Folco, qui, forte des auditions qu’elle a menées, a identifié les faiblesses de cette proposition de loi.

renforcement se ferait au détriment de la Défenseure des droits, qui dispose pourtant – cela a été dit – d’une expertise ancienne et reconnue dans la conduite de tests individuels et qui est, du fait de son indépendance, la plus à même de gérer les cas où l’administration serait responsable d’une discrimination.

femmes. Si certains points du texte sont favorablement accueillis, d’autres dispositifs, comme la création d’un comité des parties prenantes, dont la composition et les missions apparaissent mal calibrées, ont soulevé diverses réserves. Ainsi la procédure de suivi des résultats des tests a t elle été jugée trop complexe, sa durée pouvant aller jusqu’à deux ans.

Le racisme, l’intolérance et les discours de haine n’ont jamais leur place au sein de notre République et nous les condamnons évidemment avec la plus grande fermeté. Au delà de ces violences, qui constituent la partie visible de l’iceberg, des milliers de citoyennes et de citoyens deviennent victimes de discriminations multiples. Alimenté par les haines, ce poison progresse au point qu’aujourd’hui une personne sur cinq déclare avoir été victime de discrimination. Ainsi, une personne dont le prénom a une consonance maghrébine a 50 % de moins de chances d’être rappelée lorsqu’elle demande à visiter un logement. s’agit il là que de l’un des exemples les plus connus : en réalité, les discriminations se retrouvent dans une myriade de domaines, comme l’attribution des places à l’université, l’octroi d’un prêt bancaire, l’accès aux bâtiments publics, l’accès à l’emploi, le niveau de rémunération et même la surveillance de l’espace public.

Comment expliquer que le Gouvernement s’oppose à toute traçabilité des contrôles d’identité, alors même que le Conseil d’État a reconnu qu’en la matière les pratiques discriminatoires existent bel et bien ? C’est malheureusement une évidence : à l’heure actuelle, le Gouvernement ne fait pas de la lutte contre les discriminations une priorité. Nous pensons que ce rappel est utile, car c’est dans ce contexte que nous examinons aujourd’hui la proposition de loi du député du groupe Renaissance Marc Ferracci. En proposant de développer la réalisation de tests permettant d’identifier les pratiques discriminatoires, il propose d’actionner l’un des leviers disponibles. Dans la mesure où ce texte a pour ambition de protéger les citoyennes et les citoyens contre les discriminations, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires salue évidemment cette initiative. Ces tests permettraient de collecter des preuves là où les victimes ont systématiquement du mal à demander une indemnisation. Pour autant, ce texte souffre de deux défauts majeurs. Le premier défaut est institutionnel, car il est prévu que ces tests soient organisés sous l’autorité du Gouvernement. D’une part, le Gouvernement participerait ainsi à l’élaboration des tests, y compris des tests qui visent à identifier des discriminations au sein de la fonction publique.

déclarent avoir subi « des traitements inégalitaires ou des discriminations », alors qu’elles n’étaient que 14 % quelques années auparavant. Au regard de la fréquence, de l’ampleur et de la violence des discriminations, la discussion que nous avons cet après midi doit nous inviter à prendre la mesure de leurs conséquences. Il y a, au fond, une banalité de l’expérience discriminatoire pour les minorités dans notre pays. Or les discriminations sont un mal lancinant, qui fracture la société française. Malgré ce constat, trop peu d’énergie et de moyens sont déployés pour lutter contre ces discriminations.

le plus souvent consacrés à réaliser des diagnostics et des formations – évidemment nécessaires – plutôt qu’à mettre à mal les pratiques discriminatoires elles mêmes. Alors que les discriminations balafrent notre République, si peu est fait pour s’y attaquer ! Ce peu de moyens se traduit, en outre, par un non recours au droit et aux dispositifs publics de médiation par les victimes, qui, à l’instar des délégués locaux du Défenseur des droits, demeurent Si faciliter l’accès au droit est indispensable – ne serait ce qu’en faisant mieux connaître les possibilités de recours –, les dispositifs ne sont saisis qu’à la condition que les victimes aient le sentiment qu’ils peuvent aboutir et que les discriminations seront davantage punies si elles sont avérées. S’il n’existe pas de remède miracle, des sanctions plus lourdes en cas d’infractions pourraient toutefois être envisagées. Pourquoi, par ailleurs, attendre que les victimes se manifestent ? L’inspection du travail, l’inspection générale de l’éducation nationale ou l’inspection générale de la police nationale peuvent jouer un rôle actif pour prévenir les discriminations. Plus largement, c’est une transformation des pratiques institutionnelles qui apparaît indispensable face à des discriminations largement systémiques. À ce titre, la pratique du employée et défendue par la Défenseure des droits, mise en avant par ce texte est efficace, mais elle connaît des limites. Tout d’abord, ces ne permettent pas d’identifier les causes profondes des comportements discriminatoires. Comment concevoir des dispositifs appropriés pour lutter contre les discriminations si l’on en ignore les fondements ? En outre, le peut se révéler efficace à court terme, mais il ne l’est pas pour obtenir des changements structurels ni pour lutter contre le non recours au droit. Enfin, les études par ne sont pas pertinentes pour évaluer les discriminations dans tous les domaines. Par exemple, cette méthode n’est pas opportune pour les discriminations qui s’étalent dans le temps – je pense notamment au déroulement de carrière. Les demandent donc à être complétés par d’autres approches, mais aussi et surtout par des moyens importants. C’est de ce point de vue que ce texte nous semble manquer cruellement d’ambition, malgré les besoins importants en la matière. Sur cette proposition de loi, nous partageons l’avis de la Défenseure des droits

Elle est enceinte. Elle se rendra vendredi à son dix septième entretien d’embauche. Il s’appelle Sofiane. Il est étudiant ingénieur. Il se fait contrôler par la police en moyenne deux fois par semaine. Ils s’appellent Ugo et Maxime. Ils sont homosexuels. Ils se sont fait refuser l’entrée d’un restaurant. Le terrible paradoxe de ces situations, c’est qu’elles sont à la fois révoltantes, bien sûr – je crois que nous le pensons tous –, et beaucoup trop quotidiennes pour nombre de nos concitoyens. L’Observatoire des inégalités publiait, à la fin du mois de novembre 2023, son rapport sur les discriminations en France. S’il y est fait état d’une tolérance plus répandue de nos concitoyens les uns envers les autres, la situation actuelle a pourtant de quoi nous inquiéter.

En 2017 a été établie une charte sur les discriminations à l’embauche entre le ministère du travail et les entreprises, qui ne débouche sur aucune initiative. En 2018 2019, sur l’initiative de chercheurs, des sont réalisés et transmis

Ne multiplions pas les interlocuteurs et gardons une voie de recours identifiée par tous. Je pense évidemment au rôle de la Défenseure des droits, à condition, madame la ministre, qu’elle en ait réellement les moyens et que nous puissions amplifier ces derniers, notamment sur les. Pour ce qui concerne le versant méthodologique du texte, la suppression de l’article 2 visant à l’instauration d’un comité des parties prenantes ne permet plus l’intégration d’acteurs en lien direct avec les problématiques de discrimination, et fragilise la construction d’une action publique pertinente et efficace. L’article 3 manque également à la version actuelle du texte. Il nous semble essentiel qu’un test qui révèle de potentielles pratiques discriminatoires soit suivi d’effets

Les discriminations nourrissent le repli, le ressentiment et les sentiments d’injustice et d’inégalité. Elles engendrent un coût économique, qui pèse souvent lourd pour des populations déjà vulnérables. Elles entravent l’accès à l’ensemble des biens et services, y compris les services publics. Elles ont également des conséquences sociales et psychologiques importantes, prolongent des situations de détresse et amènent au renfermement social. Légiférer sur la lutte contre les discriminations est essentiel, mais ne portera des résultats probants que si la volonté du législateur est accompagnée de celle du Gouvernement pour tracer une politique publique claire et affirmée. C’est pourquoi ce texte doit être une étape, un outil supplémentaire, qui doit s’inscrire dans une ambition plus globale, « une stratégie nationale cohérente […] de lutte contre les discriminations », que la Défenseure des droits appelle de ses Un patchwork d’études statistiques apportera sans aucun doute des éclairages, mais ne constituera ni une réponse satisfaisante pour les victimes ni un outil complet pour prévenir Les violences discriminantes que vivent nombre de nos concitoyens ne sont pas acceptables dans notre République. Le groupe RDSE soutient évidemment toutes les mesures visant à lutter efficacement contre les discriminations.

Le Président de la République ne dit d’ailleurs rien d’autre lorsqu’il affirme que « faire aimer la République, c’est tenir la promesse d’émancipation qui lui est intrinsèque ». Trahir cet engagement serait se résoudre à un régime d’inégalités sociales, qui, de fait, maintiendrait les individus à leur place et nierait les aspirations légitimes de chacun. Trahir cet engagement serait se résigner à ce que certains tournent le dos à la République, qui n’aurait de République que le nom. Trahir cet engagement serait aussi, en quelque sorte, faire le lit des communautarismes et des séparatismes, contre lesquels nous combattons. En se fixant pour objectif de renforcer la lutte contre les discriminations, qui sont justement la négation du principe même d’égalité, la proposition de loi que nous examinons s’inscrit dans le prolongement de cette promesse républicaine d’émancipation. Discriminer, c’est traiter une personne de manière moins favorable qu’une autre dans une situation comparable, selon un critère qui ne justifie pas cette différence de traitement. Bien que la France dispose d’un important arsenal juridique pour lutter contre les discriminations, l’ensemble des données convergent pour confirmer leur persistance dans La Défenseure des droits indiquait ainsi avoir reçu 6 703 réclamations liées à des discriminations en 2023, contre 5 215 en 2021. Ces données démontrent l’efficacité limitée du cadre juridique en vigueur, qui ne suffit pas, à lui seul, à dissuader et à lutter efficacement contre les discriminations. Les recours contentieux constituent, en effet, des démarches lourdes à mettre en œuvre pour les victimes. Si, depuis le début des années 2000, le principe des tests est reconnu comme un outil de preuve dans le cadre d’une action en justice, force est de constater que cela ne fonctionne pas. Ainsi, en 2020, il n’y a eu aucune condamnation pénale liée à une discrimination – aucune Il y a pourtant urgence à combattre les discriminations. Comme je le soulignais en introduction, ces pratiques minent les fondements mêmes de notre pacte républicain. Elles relèguent une partie de nos concitoyens en marge de la société, en les privant de leurs droits et de leur dignité. Lorsqu’elles reviennent à priver une partie de nos concitoyens de l’accès à des biens ou à des services, elles contribuent à fragiliser encore plus des populations souvent déjà vulnérables. plus, ces pratiques représentent également un coût économique colossal pour notre pays. Selon une étude de France Stratégie réalisée en 2016, le coût économique des discriminations pourrait représenter jusqu’à 14 % de notre PIB. Dans ce contexte, la proposition de loi présentée par le député Marc Ferracci, dont je tiens à saluer l’engagement sur ce sujet important, s’inscrit dans le prolongement du Plan national de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine 2023 2026. L’ambition du texte était principalement de développer la pratique des tests individuels et statistiques, afin de mieux détecter, prévenir et corriger les discriminations dans notre pays. Si son examen par la commission a bien révélé un relatif consensus quant à l’objectif, celle ci n’a pas jugé les mesures proposées de nature à lutter efficacement contre les discriminations.

de la Défenseure des droits, la commission a supprimé toute mention des tests individuels et limité ses missions principalement à la production de tests statistiques. Le groupe RDPI regrette que la commission ait retenu une telle approche, plutôt que de voir dans la pratique des tests individuels développés par les deux institutions une potentielle complémentarité. La suppression de cette possibilité obère également toute éventuelle montée en puissance de ces tests, qui constituent pourtant un outil efficace de lutte contre les discriminations. La commission a également supprimé l’article 2, visant à créer un comité des parties prenantes, dont l’objectif aurait été de diffuser la culture des tests à l’ensemble des acteurs et, ainsi, de renforcer l’acceptabilité de cette pratique. Dénonçant son caractère correctif, elle a supprimé l’article 3, qui fournissait une base législative au, à savoir la publication des résultats des tests statistiques. Cette publication n’intervenait pourtant qu’en dernier recours, si le contrevenant manquait à définir, par le dialogue social, un plan de lutte contre les discriminations. En commission, Mme la rapporteure, dont je salue le travail, a pourtant souligné fort justement que « la lutte contre les discriminations ne [pouvait] être efficace que lorsqu’elle suscit[ait] l’adhésion des employeurs ». La proposition de

Ils redoutent surtout que, si la proposition de loi venait à être adoptée en l’état, le Sénat ne témoigne qu’une faible ambition dans la lutte contre les discriminations et, ainsi, un intérêt moindre pour la République lorsque celle ci est synonyme de promesse d’émancipation.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, dans le cadre d’un, SOS Racisme a publié ce jour même une étude dévoilant que 61 % des agences d’intérim acceptaient de faire une présélection des candidats en fonction de la couleur de leur peau. Aujourd’hui, en France, les candidats ayant un nom d’origine française ont près de 50 % de chances de plus d’être rappelés par un recruteur que ceux qui ont un nom d’origine maghrébine.

les candidats dont le nom était d’origine française ont été rappelés dans 33,3 % des cas par les employeurs, contre 22,8 % pour ceux ayant un nom d’origine maghrébine. En 2022, en France, selon l’Insee, seules 44 % des personnes en situation de handicap étaient actives, contre 75 % de l’ensemble de la population. Aujourd’hui, en France, le fait de porter un nom de famille d’origine maghrébine ou d’Afrique de l’Ouest réduit fortement la probabilité d’obtenir une visite pour louer un appartement. Dans le cadre d’une opération de réalisée en 2016

avec une candidature tout à fait semblable – en termes d’emploi, d’âge et de nationalité –, le candidat d’origine maghrébine n’a reçu que 10,1 % de réponses positives et le candidat d’Afrique subsaharienne seulement 9,4 %. Le candidat Le candidat au nom français avait donc 1,5 fois plus de chances que le candidat originaire d’Afrique subsaharienne de visiter ce logement. Aujourd’hui, en France, les jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes ont une probabilité vingt fois plus élevée que les autres d’être contrôlés par les forces de l’ordre, selon une étude du Défenseur des droits publiée en 2017. La Défenseure des droits a indiqué avoir reçu 6 703 réclamations liées à des discriminations en 2023, contre 5 215 en 2021. Les trois principales causes de discrimination sont le handicap – 21 % –, l’origine – 13 % – et l’état de santé – 9 %. Aujourd’hui, en France, nous devons donc nous résoudre à reconnaître que de nombreux concitoyens sont confrontés à la violence des discriminations chaque jour, dans leur vie quotidienne. Cette situation n’est pas acceptable. Elle remet en cause le principe d’égalité, qui est le fondement de notre pacte républicain. Elle alimente un ressentiment légitime chez de nombreux Français et met à mal notre vivre ensemble. Bien évidemment, il faudra bien plus qu’une simple proposition de loi visant à développer les tests individuels et statistiques afin de mettre fin aux discriminations structurelles qui rongent notre République Il nous faudra un sursaut collectif, une prise de conscience et, surtout, une volonté de mettre fin à ces pratiques discriminatoires. Aujourd’hui, cette proposition de loi prévoit de confier à un service placé sous l’autorité du Premier ministre la réalisation de tests de discrimination individuels et statistiques.

Bien sûr, nous souscrivons à l’objectif du texte. En revanche, ses modalités soulèvent de nombreuses interrogations. Premièrement, l’article 1 prévoit de confier à la Dilcrah une compétence élargie en matière de prévention et de correction des situations de discrimination, avec la réalisation de tests individuels et statistiques.

Dans son avis, la Défenseure des droits, qui salue le sens du texte, se dit néanmoins clairement défavorable à l’idée de confier de telles compétences à un service de l’État qui ne présente aucune garantie d’indépendance.

et reconnue dans la réalisation de ces tests. Elle est la plus compétente pour accompagner les victimes de discriminations sur la voie judiciaire, en particulier si l’auteur des discriminations est une administration. Nous saluons les modifications apportées en commission sur l’initiative de Mme la rapporteure : elles vont dans le bon sens. Nous souhaitons, en revanche, rétablir l’objectif d’œuvrer « à la correction des situations de discrimination, notamment en matière d’accès à l’emploi, au logement et aux biens et services publics ou privés viens à l’article 2, qui créait un comité des parties prenantes. L’effectif de cet organe n’était pas clairement défini et les modalités de nomination de ses membres étaient renvoyées à un décret en Conseil d’État, laissant le flou sur leur nomination, donc leur indépendance. Nous saluons également la suppression de cet article en commission. quant à lui, la procédure applicable lorsqu’un test statistique révèle des pratiques discriminatoires. Madame la rapporteure, vous avez choisi de supprimer purement et simplement cet article. Nous considérons que c’est un problème. Évidemment, cet article n’était pas parfait, mais que vaut un texte visant à lutter contre les discriminations dénué de toute sanction ? Rien. La sanction prévue était déjà très légère pour la personne morale concernée. Vous semblez considérer que les entreprises sont toutes de bonne volonté et prêtes à cesser leurs discriminations un dialogue informel… C’est malheureusement bien trop idéaliste et éloigné de la réalité et de la pratique Bien sûr, un nombre croissant d’entreprises prennent volontairement des mesures pour corriger les biais discriminatoires dans leurs pratiques, parce qu’elles prennent à cœur leur responsabilité sociale ou, plus pragmatiquement, parce qu’elles prennent au sérieux les nombreuses études démontrant que la diversité des ressources humaines est un facteur de réussite économique. Malheureusement, beaucoup d’autres entités – personnes morales privées ou publiques – n’agissent que si elles y sont contraintes ! Si le droit existant suffisait, les discriminations relèveraient aujourd’hui de l’exception aberrante. Nous savons bien que la réalité est tout autre. Force est de constater que la pratique du fonctionne. Elle permet de mettre la pression en amont sur les entreprises, qui développeront leurs bonnes pratiques par peur d’une atteinte à leur réputation. Elle est efficace dans plusieurs domaines. Aussi proposerons nous de rétablir l’article 3, en prévoyant, en plus, que le procureur de la République soit informé des infractions constatées et que le montant de l’amende administrative passe de 1 % à 5 % des rémunérations et gains. Nous proposerons également une interdiction complémentaire de candidater aux marchés publics pour les entreprises épinglées qui n’ont pas pris de mesures suffisantes. Madame la ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, vous l’aurez compris, l’objectif de ce texte est louable : il s’agit de mieux lutter contre les discriminations. Ces discriminations étant structurelles dans notre pays, il faudra également mieux lutter contre les stéréotypes et les préjugés, ce qui nécessite des mesures bien plus ambitieuses. Je me joins à Mme la rapporteure pour appeler l’attention du Gouvernement sur l’importance de créer un observatoire indépendant des discriminations. De notre côté, nous ne voterons cette proposition de loi que si nos amendements visant à améliorer les dispositifs et à assurer une meilleure indépendance des acteurs chargés de lutter contre les discriminations sont adoptés.

Initialement, cette proposition de loi visait à généraliser la pratique du pour lutter contre les discriminations, notamment dans l’accès à l’emploi, au logement, aux prêts bancaires ou aux services publics.

des potentielles victimes, alors que celui ci a désormais acquis une certaine notoriété auprès de nos concitoyens. Nous saluons donc la suppression de la référence aux tests individuels par notre rapporteur. En outre, la création d’un énième comité à l’article 2, le comité des parties prenantes, n’est pas satisfaisante. Sur ce point, rien ne remplace le rôle des pouvoirs publics et le dialogue social conduit par les partenaires sociaux Par ailleurs, nous ne mesurons pas non plus la pertinence de la procédure prévue à l’article 3, lorsque le résultat d’un test statistique révèle de potentielles pratiques discriminatoires. Faire intervenir successivement la Dilcrah, le comité des parties prenantes, les partenaires sociaux et l’administration du travail prendrait des mois, pour des résultats pour le moins incertains,

Au delà de la technicité de ces diverses mesures, je souhaite élargir mon propos en y ajoutant quelques éléments de contexte. En France, aujourd’hui, les entreprises peinent à embaucher. Je vous rappelle, mes chers collègues, que, si les entreprises rencontraient déjà des problèmes de recrutement en 2022 et en 2023, ceux ci continuent de s’accroître en 2024, quelle que soit la taille de l’établissement

des entreprises qui pratiquent de plus en plus l’auto ? Notre rôle, comme celui des pouvoirs publics, n’est il pas d’encourager ces initiatives, d’accompagner les comportements vertueux, plutôt que de menacer de faillite

toutes les discriminations qui découlent de ces derniers. Il est donc impératif que les tests statistiques permettent d’engager des mesures de correction. Par ailleurs, nous souhaitons rétablir

Cette précision, qui peut paraître superfétatoire, est d’une grande importance symbolique. Je rappelle que le rapport de l’Observatoire des inégalités de la fin de 2023 démontrait que l’origine était

fin, l’amendement prévoit donc de rétablir une disposition qui a été adoptée en séance publique à l’Assemblée nationale, mais supprimée par la suite.

commission a estimé que la compétence de la Dilcrah devait se limiter à la réalisation des tests et qu’il revenait à l’administration du travail d’accompagner l’organisation dans la transformation de ses pratiques. J’en viens à

pas forcément aujourd’hui. J’insiste également sur le fait que les discriminations à l’emploi et à l’embauche sont bien évidemment couvertes par le terme générique retenu pour notre rédaction. De même, tous les services sont couverts, privés comme publics. L’avis est donc défavorable sur ces trois amendements.

des outils statistiques, ni plus ni moins. Les réaliser sur de trop petites organisations serait donc probablement inutile. Les résultats obtenus seraient trop précaires pour tirer des conclusions définitives sur la conformité des pratiques de l’organisation en matière de discrimination. Il est donc logique d’imposer une limite. Quel est l’avis

avoir un impact sur le choix des organismes à tester, la méthodologie ou les conséquences à donner aux tests. Ces situations délicates pourraient malheureusement survenir assez fréquemment. On peut penser à la fonction publique, mais aussi aux entreprises détenues ou contrôlées par l’État, qui emploient 3,1 % des salariés en France. Quand un test de discrimination vise l’une de ces entreprises, l’État n’est pas neutre. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons confier la définition des orientations au Défenseur des droits,

ai renoncé ! Enfin, la solution que vous proposez présente à mon sens un défaut important. Elle fait de la Dilcrah un sous traitant du Défenseur des droits. Or il ne revient pas à une autorité indépendante de dicter le programme de travail d’une administration de l’État,

: nul besoin de se cacher derrière des artifices statistiques quand on veut voter contre un texte, il faut assumer

pas jugé opportun d’inclure les organisations syndicales dans la définition des orientations des tests et des suites qu’il convient de leur donner. Avait été ainsi créé un comité des parties prenantes, dont il n’était pas prévu qu’il soit ouvert aux syndicats. Or les organisations syndicales nous semblent disposer d’une expertise en la matière et être capables de conseiller les travailleuses et les travailleurs qui s’estiment victimes de discrimination.

ou en militant pour des actions de groupe. C’est pourquoi notre amendement prévoit que les syndicats et les associations de lutte contre les discriminations puissent participer à l’élaboration des orientations guidant les tests.

Un système de reconnaissance vocale permettant le pilotage d’hélicoptères est difficilement utilisable par des femmes, car son algorithme est programmé pour la seule reconnaissance des voix masculines – apparemment, une femme ne peut pas piloter un hélicoptère. La marge

Néanmoins, il ne semble pas que la voie que vous proposez permette en pratique de répondre efficacement à ce cas de figure. Premièrement, la Dilcrah ne dispose pas des compétences techniques pour procéder à l’analyse du code source

cherchant à recruter des travailleurs « de préférence européens, idéalement caucasiens ». C’était un peu piégeux, je vous le concède… Résultat : dans 61 % des cas,

est à M. Guy Benarroche. Nous devons sanctionner toutes les discriminations de la même manière, peu importe le mécanisme qui les sous tend. Il en est de même pour les algorithmes – j’y reviens. De nombreuses études ont démontré que les algorithmes, par exemple ceux qui sont utilisés pour la reconnaissance faciale, reproduisent les discriminations issues des biais de leurs programmeurs.

Pour mettre un terme à ces pratiques, nous demandons de réprimer le recours à un algorithme dont le fonctionnement discriminatoire a été révélé par un test, dans le prolongement des infractions déjà prévues par le code pénal.

Je comprends votre intention, mais le dispositif ne me semble pas applicable en l’état. En effet, pourquoi lier la sanction à la publication des résultats d’un test de discrimination ? Dans certains cas, l’employeur pourrait avoir pris connaissance des biais de l’algorithme

aux personnes morales publiques ou privées comptant plus de 1 000 employés rend cette proposition de loi vraiment mauvaise, donc totalement indéfendable. En conséquence, nous voterons contre l’ensemble du texte.

n° 154 : Le Sénat a adopté. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant diverses mesures relatives au grand âge et à l’autonomie est parvenue à l’adoption d’un texte commun.